parole est à Monsieur Daniel Breuiller en 1er, rapporteur spécial de la commission des finances pour sept minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame et messieurs les rapporteurs, chers collègues, avec plus de 20 milliards d'euros, la mission Travail emploi est après la mission écologique, celle dont la progression est la plus forte par rapport à la loi de finances initiale 2022 cependant, compte tenu du volume très important de crédits supplémentaires provenant 21 et 22 de collectif budgétaire du plan de relance et de fonds de concours, nous serons en réalité dans des ordres de grandeur comparable à ceux constatés ces 2 dernières années, ces mouvements en cours d'exercice et les écarts considérables entre crédits votés et exécuté ont notablement brouiller la lisibilité du budget de l'emploi et de la formation professionnelle depuis 2 ans, nous espérons nous prononcer aujourd'hui sur des bases plus conforme à ce que sera réellement l'impact de ce budget en 2023, j'évoquerai plus particules plus particulièrement le volet de la mission relatifs à la politique de l'emploi tout d'abord je voudrais dire que les moyens très important consacré depuis 2020 à la politique portée par cette mission ont certainement joué un rôle dans l'amélioration de la situation de l'emploi, je pense notamment à l'apprentissage, la hausse du nombre de contrats d'apprentissage représentent près de la moitié de la baisse du nombre de chômeurs, la dépense budgétaire s'est alourdi d'autres dépenses ont diminué et l'assurance chômage n'est plus en déficit concernant la mission, le recul du chômage entraîne une nette diminution des dépenses d'allocations, prise en charge par l'État, de l'ordre de 500 millions inversement la progression de l'emploi, major de près de 700 millions la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations, il s'agit d'une dépense qui atteint 5 milliards d'euros, soit un quart du budget total de la mission, s'agissant des actions en faveur de publics spécifiques, le budget destiné aux entreprises adaptées, poursuit sa progression, le contrôle effectué par Emmanuel Capus pour la commission des finances montre plusieurs freins subsistant développement de ce type d'emploi d'expérimentation de nouvelles formes d'insertion dans l'emploi des personnes handicapées, n'a pas encore donné les résultats escomptés, les dotations pour l'insertion par l'activité économique sont maintenus au niveau de 2022, ce qui diminuera le nombre d'emplois finançable, elles ont certes notablement augmenté depuis 3 ans, mais cette simple stabilisation pose question : les rémunérations des bénéficiaires de l'IAE indexé sur le SMIC vont augmenter à crédit égaux, il pourrait donc avoir moins de bénéficiaires, les acteurs de l'IA, manque de visibilité sur la répartition territoriale de l'enveloppe entre les différents types de structures alors que le coût des contrats sera plus élevé, les actions en faveur de l'accompagnement renforcé des jeunes vers l'emploi prennent quant elle une part accrue dans le budget de la mission avec le contrat d'engagement jeune CEJ mis en place le 1er mars dernier et dont la dotation atteint un milliard d'euros, ce dispositif a été introduit dans des conditions critiquables sans évaluation préalable en cours de discussion budgétaire du PLF 2022 le recul manque pour en effectuer une évaluation approfondie, toutefois, les premiers éléments recueillis sont plutôt encourageants sa montée en charge, objectif 300000 jeunes cette année concernera essentiellement les missions locales, sur lesquelles repose en majorité cet accompagnement intensif des jeunes présentant comme on dit pudiquement des besoins périphérique important l'état leur apporte un soutien sensiblement supérieure, je parle des missions locales à celui dont elle bénéficiait il y a encore 3 ou 4 ans, des conditions d'orientation des jeunes soit vers Pôle Emploi, soit vers les missions locales ont été clarifiées, il semble que le CO et même permis d'améliorer les échanges entre 2 opérateurs agissant jusqu'à présent de manière trop cloisonné, la gestion du dispositif pourrait induire une charge administrative assez lourde au détriment des charges d'accompagnement notamment pour satisfaire aux conditions d'activité minimale, il y a sans doute matière à simplifier dans ce domaine, de même, il faudra être vigilant pour que le CE s'articule au mieux avec les structures comme les écoles de la 2ème, chance ou des en résumé le CSJ me paraît améliorer le dispositif de la garantie, jeunes et mérite d'être consolidé, j'ai mentionné pour l'emploi, la subvention de l'État avait baissé jusqu'en 2021 elle a été stabilisé en 2000 22 et augmente de 136 millions en 2023 dans le même temps, les crédits attribués au au titre de la mission, plan de relance ne sont pas reconduits, le plafond d'emplois de Pôle emploi en très légère baisse sera globalement maintenue en 2000 23 au niveau de ces 2 dernières années, ces moyens ont été renforcées pour le CEJ l'accompagnement des chômeurs de très longue durée et le plan de réduction des tensions de recrutement toutefois les évolutions de Pôle emploi au au-delà de 2023 sont suspendus aux résultats des travaux lancés sur France travaille le gouvernement, Monsieur le Ministre, s'est défendu de vouloir fusionner au refondre l'organisation des acteurs du service public de l'emploi, pour autant, à ce jour, vous n'avez pas indiqué en quoi consistera cette réforme, on nous a plutôt dit en quoi elle ne consisterait pas à mon sens l'enjeu porte sur une réelle coordination des acteurs de terrain pour mieux identifier les personnes nécessitant un accompagnement mieux orienter mieux partager des données mieux assurer de suivi, je ne sais à ce stade-ci France répondra réellement à ce besoin, je relève que les prévisions indicatif pour les dépenses de fonctionnement du programme accès retour à l'emploi, constitué à près de 90 % de la subvention à Pôle Emploi marque une diminution de 11 % en 2000 vingt-quatre et de 12 % en 2025, le recul du chômage ne doit pas masquer la persistance d'un nombre encore bien trop important de personnes très éloignées de l'emploi, notamment parmi les jeunes, c'est pour ces publics que les besoins d'accompagnement, ce sont les plus élevés, l'effort en leur direction doit être maintenue et même renforcée pour les mêmes raisons, je suis attaché à ce qu'en matière d'apprentissage et de formation professionnelle, une attention prioritaire soit porté à ceux qui ont le moins de facilité à s'insérer sur le marché du travail ou à accéder aux formations, voilà les observations que je souhaitais formulées sur cette mission en mon nom et en mon nom et en celui de mon co-rapporteur, Emmanuel Capus, mission dont les crédits sont confortés dans ce projet de budget la commission des finances suivant sagement nos recommandations, vous en propose l'adoption. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à monsieur Emmanuel Capus. Rapporteur spécial également de la commission des finances. également pour cette minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais donc pour ma part, aborder le second volet de la mission, à savoir le financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, le succès de l'apprentissage, au-delà de toute prévision et paradoxalement la source d'une des difficultés budgétaires majeures de cette mission avec un poids financier qui dépasse largement celui de toutes les autres missions, pardon, c'est un sujet d'inquiétude exprimée à de multiples reprises en commission comme en séance publique, particulièrement à l'occasion des rallonges budgétaires successives accordée à France compétences ces inquiétudes sont légitimes mais l'apprentissage comme la formation professionnelle constitue aussi un enjeu essentiel si nous voulons progresser vers le plein emploi un objectif vers lequel beaucoup de chemin reste à parcourir, même si la situation s'est améliorée, puisque par rapport à fin 2019, l'emploi salarié a progressé de 800000 personnes et le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de près de 400000 personnes. Présenté de longue date comme la meilleure voie d'insertion professionnelle des jeunes, l'apprentissage a longtemps stagné. Le nombre annuel de contrats conclus a même baissé de 2012 à 2017 avant de remonter nettement en 2018 et 2019 puis de décoller à un rythme tout à fait inattendu près de 740000 contrats conclus en 2021 2 fois plus qu'en 2000 19 et autant, sinon plus, en 2022. Sous l'angle budgétaire la question de l'apprentissage se pose à 2 niveaux assez différent, le 1er est celui du soutien de l'État à travers les aides à l'embauche. L'aide exceptionnelle mise en place en 2020, qui concerne toutes les entreprises, y compris les entreprises de plus de 250 salariés et les formations allant jusqu'au bac plus cinq a certainement joué dans l'essor de l'apprentissage, mais le coût budgétaire a bondi de 1,3 milliards en 2020 à 4 2 milliards en 2021 pour 2022 le montant sera certainement du même ordre, la question d'un nouveau paramétrage de cette aide est aujourd'hui posée, elle fait l'objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ce qui me paraît tout à fait approprié, il est certainement nécessaire de faire la part entre 2 probable effet d'aubaine et les incitations utiles au maintien de la dynamique actuelle de l'apprentissage, il semble exclu de revenir purement et simplement à l'aide unique d'avant 2020, mais nous ignorons pour l'heure, si l'on s'oriente vers une diminution du montant de l'aide actuelle ou un ciblage sur certaines entreprises ou certains niveaux de formation peut-être Monsieur le Ministre, serez-vous en mesure de donner quelques indications sur les options privilégiées. Et Madame la Ministre, également, en tout état de cause, tous les contrats conclus avant la fin de l'année 2022 bénéficieront pour un an de l'actuel régime des aides à l'embauche, l'effet budgétaire d'une révision à la baisse ne se fera donc sentir qu'à l'échéance des contrats actuels et à la conclusion de de nouveaux contrats, c'est-à-dire en large partie sur les 4 derniers mois de 2023, c'est la raison pour laquelle un amendement de réduction de crédits me paraît pas nécessairement efficace mais c'est surtout la situation financière de France compétences qui pose le problème budgétaire le plus difficile, l'État a dû intervenir à hauteur de près de 3 milliards en 2021, puis à nouveau de 4 milliards en 2022, ce qui n'évitera pas un déficit estimé autour de 3 milliards et demi en fin d'année. Je rappelle qu'à sa création, aucun soutien de l'État, cet opérateur n'a été envisagée, à l'inverse, la loi de 2018 prévoit même le versement à l'État par France compétence d'une contribution à la formation des demandeurs d'emploi, contribution de 1 virgule 6 milliards d'euros par an depuis 2019, l'écart s'est rapidement creusé entre les ressources de France compétences qui évolue en fonction de la masse salariale et ses dépenses, à savoir le financement de l'alternance et celui du CPF, ces 2 dispositifs constituant des enveloppes ouvertes. S'agissant plus particulièrement du CPF, qui représente environ un 5ème des dépenses un certain nombre de mesures de lutte contre la fraude de sécurisation de déréférencement d'organismes ont été prises. Des dispositions législatives figure dans la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale qui sera discutée ici même le 8 décembre prochain le très large éventail de formations finançable rend nécessaire incontestablement une régulation dont le principe a été introduit dans l'article 49 rattachés à la mission, je soutiens ce principe et je proposerais de le préciser, par un amendement que nous examinerons tout à l'heure par ailleurs à travers le projet de loi de finances, l'État des charges France compétence d'une bonne part de la contribution qu'elle lui verse au titre de la formation des demandeurs d'emploi, comme l'a souligné la Cour des comptes, le niveau de cette contribution paraissait excessif d'autant plus que les dotations du pic qu'elle vient abonder ne sont que partiellement et font l'objet de report important. Deuxièmement, une subvention à France compétences d'un montant de 1,7 milliard est inscrite d'emblée dans les crédits de la mission de ce point de vue le PLF 2023 m'apparaît plus sincère que celui de 1022 qui passait totalement sous silence ce déficit, l'ensemble de ces mesures atténue la contrainte financière sur France compétences sans pour autant, nous le savons bien son équilibre financier, une révision des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage est intervenu en septembre dernier avec un effet l'économie évaluée à 200 millions en 2023, une autre révision doit intervenir en avril 2023 au-delà il faudra sans doute définir des priorités en terme de niveau de soutien selon les différents types de structures et le niveau de formation. L'image de l'apprentissage s'est profondément transformé, c'est un acquis majeur de la réforme qu'il faut préserver, mais il est maintenant indispensable que l'État en lien avec les partenaires sociaux. Et définissent une trajectoire soutenable pour les financements de la formation professionnelle et de l'apprentissage sans casser la dynamique en cours, c'est la raison pour laquelle mes chers collègues sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances vous propose. Comme l'a dit mon collègue, co-rapporteur Daniel Breuiller l'adoption des crédits de la mission Travail et emploi pour 2023. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à madame Puissat, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour 2023 la mission Travail emploi se caractérise par une progression considérable de ses crédits plus plus 42 % et par de nombreuses incertitudes le devant de prononcer alors que de nombreux changements sont attendus en 2023 lancements de France travaille redéfinition des aides à l'apprentissage fait attendu du pic financement toujours de France compétences dans ce contexte, la commission des affaires sociales propose de diminuer les crédits de cette mission sur 2 postes de dépenses la subvention à France compétences et le pic si on veut continuer de développer l'apprentissage et la formation professionnelle, il est urgent de sécuriser leur financement, or, à ce stade, aucune réponse pérenne est apporté au déséquilibre financier de France compétences l'établissement, accumule les déficits, alors même qu'il va recevoir 4 milliards d'euros de subventions en 2 1000 22 et qu'une enveloppe de 1,6 milliards d'euros, est prévue pour 2023, il est urgent de régler cette situation aujourd'hui insoutenable de premières mesures de régulation des dépenses sont engagés, il faut aller plus loin en proposant à cet effet d'instituer un plafonnement de la prise en charge par le CSP du coup de certaines formations, amendement qui a été évoqué par mon collègue dans cette logique, la commission propose également de diminuer de 300 millions d'euros, la subvention à France compétences cette réduction doit être la contrepartie d'une plus forte régulation des dépenses d'apprentissage et du CPF et d'une réduction plus significative de la contribution de France compétences au pic concernant le pic qui a été prolongée jusqu'en 2023, nous pensons que l'année prochaine devrait être marquée par une revue des dispositifs financés par ce plan afin d'évaluer l'opportunité de maintenir leur financement à ce stade, les annonces du gouvernement, non ça n'ont pas apporté de précisions sur l'avenir de ces dispositifs, ni même sur la fin effective du pic sans affecter le développement de la formation dans les régions ne semble qu'une telle évaluation doit être rapidement engagé et que les moyens du pic doivent correspondre à ceux d'une dernière année d'exécution, considérant que ce plan doit prendre fin prochainement que sa contribution directe à la formation et l'insertion n'est pas mesuré et que son pilotage et toujours pas satisfaisant, nous proposons de diminuer les moyens du pic à hauteur de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement s'il faut se réjouir de la diminution des dépenses d'allocations de solidarité pour les demandeurs d'emploi, signe d'une conjoncture favorable, le luxe avons pas de corrélation dans les moyens alloués à Pôle Emploi qui, eux, progressent de 17 % il faudra sans tarder, évaluer la pertinence du maintien des effectifs de Pôle Emploi qui avaient été accordés à titre exceptionnel, lors de la crise sanitaire en matière d'insertion dans l'emploi, la réduction des objectifs d'entrées en contrat aidé et en emplois francs paraît adapté à l'amélioration de la situation de l'emploi, la trajectoire de montée en charge du contrat d'engagement jeune est également cohérente, il faudra mesurer les effets de ces dispositifs sur l'insertion dans l'emploi durable en particulier dans le cas de la mise en place de France travaille sous réserve de ces observations, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission et aux articles qui sont rattachés voici monsieur le Président, 3 minutes d'intervention qui peuvent rapporter gros pour le budget de l'État, je vous remercie. Pardon. Il reste même dix secondes à la suite de notre discussion, je rappelle que le temps de parole autorisée à chaque groupe pour chacune des discussions qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote il n'y a pas de duplication, par ailleurs, le gouvernement dispose au total, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, de 15 minutes pour intervenir, nous commençons donc la discussion générale proprement dite, la parole est à Bernard Jomier pour 9 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la mission Travail emploi pour 2023 s'élève à vingt milliards 900 millions d'euros si la progression de ce budget par rapport à 2022 semble importante, il fait ce qu'on vient de là, relativiser en effet ces chiffre sont le résultat d'une plus grande compensation des exonérations de cotisations sociales compensations qui représentent à présent un quart des crédits de la mission mais aussi cette hausse affichée des crédits résulte de changement de périmètre certains dispositifs étant financé l'an prochain par le budget du ministère du Travail, après avoir été pris en charge jusque fin 2022 par des crédits du plan de relance au final ah bien Inès regarder l'exercice 2023 débutera avec un niveau de crédit proche de l'an dernier et l'avenir n'est pas rigueur puisque le gouvernement a déjà acté une baisse importante du budget de la mission, pour 2024 et 2025, il ne s'agit pas évidemment de nier que le taux de chômage s'élève à 7 4 % à la fin du second trimestre, mais nous voulons rappeler que l'OFCE prévoit une remontée du nombre de demandeurs d'emploi en 2023 et 2024 et surtout gardons à l'esprit que nos concitoyens les plus éloignées du marché du travail sont ceux pour lesquels les freins préalable au retour à l'emploi sont nombreux, il est donc indispensable que les politiques publiques soient adaptée pour mieux prendre en charge ceux pour qui les obstacles semblent parfois insurmontable, il y aurait beaucoup à dire sur notre marché du travail, tout d'abord parce que la semaine dernière, nous avons eu la confirmation dans le rapport annuel le Proxinvest que les rémunérations des dirigeants des 120 plus grandes sociétés cotées ont augmenté en moyenne de 22 % par rapport à 2019 portant la rémunération moyenne à 4,5 millions d'euros, c'est un record historique depuis 15 ans. Et le même jour, quasiment, vous, monsieur le ministre du Travail, vous présentiez les nouvelles règles d'assurance chômage à niveau en défaveur des plus fragiles et des seniors, il faut rappeler que seuls 55 % des 55 64 ans travaillent dans notre pays et que ce taux d'emploi reste de 6 points inférieurs à la moyenne des pays européens, malgré ces constat largement partagé : le gouvernement a choisi de réduire de 25 % la durée d'indemnisation pour tous les salariés en fin d'indemnisation et nouvellement inscrits à Pôle Emploi à compter du 1er février prochain, ce sont ainsi près de 3 à 4 milliards d'euros d'économies qui seront réalisées au détriment des salariés et des chômeurs, et nous considérons que ce n'est pas acceptable l'idée selon laquelle une baisse des droits des demandeurs d'emploi, améliorer leur entrée sur le marché du travail est un leurre, les difficultés de recrutement actuel vient d'abord d'un déficit de compétences qui, aux besoins des entreprises et également des conditions de travail proposé, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne souscrivons pas à l'idée selon laquelle il faudrait donner toujours moins allocataires indemnisés par l'assurance chômage et affaiblir encore davantage le service public de l'emploi, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il est toujours plus difficile d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller Pôle Emploi : les délais sont d'autant plus important d'ailleurs que les horaires d'accueil sont réduits, on demande aux aux aux allocataires de se débrouiller seuls face à leur ordinateur en somme de faire leurs démarches en ligne, ce qui occasionne de réelles difficultés pour nombre d'entre eux, car rien ne remplace un accueil physique par un professionnel formé et à l'écoute, le résultat d'ailleurs, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de contestation pour cause d'erreurs dans le calcul des indemnités notamment, il n'y a jamais eu autant de conseillers agresser verbalement ou, pire, tant les tensions sont importantes et nous doutons que les choses aillent mieux avec la nouvelle réforme qui va apporter encore de la complexité et accroître les incompréhensions, j'entends le gouvernement nous expliquer qu'il faudrait faire des économies, mais je réponds qu'avec un dans un budget, pardon, ce sont des dépenses mais aussi des recettes et que les choix opérés aujourd'hui sont avant tout, évidemment, des choix politiques depuis l'ouverture des débats sur le PLF et auparavant sur le PLFSS notre groupe a formulé de nos nombreuses propositions en matière de recettes que le gouvernement rejette toute au final qui va être impacté toujours les mêmes, les plus fragiles, ceux qui subissent les contrats précaires et les périodes d'inactivité, je l'ai déjà mentionné un quart des crédits de la mission se résume à des compensations d'exonérations de cotisations sociales, nous pensons que leur impact mériterait d'être mieux évaluer d'autant plus que ces politiques s'inscrivent dans la durée car tout cela, finalement, ça coûte cher, ça coûte cher, soit la sécurité sociale soit au budget de l'État et au total, c'est un désarmement fiscal qui n'est pas sans conséquences s'agissant de l'insertion par la vie, l'activité économique qui apporte une contribution réelle à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, nous ferons des propositions si ce secteur a bénéficié d'un soutien ces dernières années, employant aujourd'hui près de 100 150000 salariés, nous ne pouvons passer l'inquiétude des parties prenantes, en raison de la hausse du SMIC sur lesquels les rémunérations des bénéficiaires de l'IAE son index on peut craindre qu'à enveloppe constante, le nombre de postes finançable soient moindres, ce qui remettrait en cause l'élan constaté le secteur regroupe par ailleurs des structures de statuts différents des entreprises intermédiaires des associations intermédiaires, des ateliers, des chantiers d'insertion avec de force d'écart d'aide au poste, les acteurs de l'IAE souligne un certain manque de visibilité pour 2023 due aux incertitudes sur la répartition territoriale de l'enveloppe entre les différents types de structures alors que le coût des contrats lui sera plus élevée qu'en 2022 concernant France compétences, je rappelle que la commission des affaires sociales a adopté au mois de juin dernier un rapport très complet intitulé France compétences face à une crise de croissance, donc Corinne Ferré, été corapporteur avec Martin lévrier et Frédérique Puissat ce rapport avait formulé 40 propositions pour une meilleure régulation CPF que de l'apprentissage, là encore, personne ne peut ignorer que dès 2020 France compétences s'est trouvé dans une situation financière très déséquilibrée, occasionnant un important déficit ce déficit à des causes structurelles dont les conséquences auraient pu être mieux anticiper, en pratique, les 2 principaux dispositifs financés par France compétence l'apprentissage et le CPF constituent des enveloppes ouvertes ainsi le nombre de places en CFA n'est plus contingentés chaque contrat d'apprentissage ou droit à une prise en charge sur les fonds de France compétences quant au droit de la formation profite désormais monétiser, ils peuvent être directement mobilisés par les titulaires du CPF avec tous les excès, dont nous discuterons d'ailleurs prochainement dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi pour faire face, des subventions au titre du soutien à la trésorerie de France compétents sont inscrites au budget sont inscrites au budget 2023, nous avions déjà cet été lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2022 acté un soutien à cette instance encore renforcer ce mois-ci par une nouvelle subvention de l'État à hauteur de 2 milliards plus globalement, on voit bien que rien ne pourra se faire sans une plus grande responsabilisation mobilisation des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui passe par un dialogue renforcé avec les branches professionnelles, avec les partenaires sociaux, il n'appartient pas au Parlement, ni au pouvoir réglementaire de se substituer à ces derniers et de faire passer les réformes certes nécessaire, mais là en force, je terminerai en soulignant que l'examen de cette mission intervient dans un contexte de préfiguration encore très floue de la réforme du service public du travail avec la création de France travail censé faire le pendant à France compétences compte tenu de ce qu'il s'est passé avec cette instance de gouvernance nationale nous émettons des craintes et nous réaffirmons notre souhait d'une meilleure coordination des acteurs de l'emploi sur le terrain pour mieux cibler, mieux identifier les personnes nécessitant un accompagnement les orienter mieux partager les données et assurer un meilleur suivi, vous vous en doutez, dans la mesure où ce budget, acte d'une réduction des dépenses du programme 102, dans la mesure où le compte n'y est pas davantage, concernant la jeunesse. Nous, notre groupe plus que j'ai un opposé à toutes les coupes budgétaires ah ces dispositifs et que vous nous vantez fondée je cite sur des droits et devoirs, alors qu'il procède d'une volonté unique de l'État, nous n'approuvons pas les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci, cher collègue, et la parole maintenant à Madame Katia pour se polie pour le groupe CRCE. Et pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation des crédits de la mission Travail, emploi de 4 à 5 milliards d'euros, cette augmentation masque en réalité une modification de périmètre de la mission avec l'intégration des crédits de l'activité partielle qui figurait auparavant dans la mission, plan de relance cette augmentation masque également la baisse des crédits destinés au programme accès et retour à l'emploi et notamment de l'indemnisation des demandeurs d'emploi de 500 millions d'euros, le gouvernement justifie cette diminution des crédits par l'amélioration de la situation de l'emploi et des conséquences de la réforme de l'assurance chômage, avec cette réforme, si le taux de chômage passe sous la barre de 9 % après une période de 6 mois la durée d'indemnisation sera réduite de 25 concrètement à partir du 1er février 2023, un salarié de moins de 53 ans ne sera indemnisé que pendant 18 mois au lieu de 24, aujourd'hui un salarié de plus de 55 ans sera indemnisée pendant 27 mois au lieu de 36 aujourd'hui, cette réforme va baisser les droits des chômeurs et, selon le secrétaire national de la CFDT n'aura pas d'effet sur l'emploi, sauf à brosser dans le sens du poil un électorat et à faire des économies budgétaires, le gouvernement veut en réalité faire 4 milliards d'euros d'économies sur le système d'assurance chômage les personnes sans emploi seront contraints d'accepter des métiers pénibles, mal payés, en réduisant les uns démission les s'indemnisation chômage, à l'opposé du projet de du gouvernement, nous considérons qu'il faut revaloriser le travail, lui redonner tout son sens, afin que chacun y retrouve le goût avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail, d'augmentation d'augmenter les salaires et de revaloriser le métier essentiel c'est vous qui portez la responsabilité de la dévalorisation du sens du travail qui n'est plus un lieu d'épanouissement mais de ma lettre et de souffrance, ce projet de loi de finances pour 2023 prévoit également la réforme du service public de l'emploi avec le projet France travail dont les contours demeurent encore très flou, si un préfet figure Aalter a été nommé pour préparer sa mise en place dès 2024, les acteurs ne dispose d'aucun élément précis sur son périmètre et son contenu, les enjeux sont multiples ainsi cuites des jeunes les plus éloignés du travail qui doivent être mobilisées affronte des problématiques dites périphériques aucun financement n'est aujourd'hui fléché vers des solutions et les missions locales ont trop peu de levier enfin, s'agissant de l'inspection du travail, nous alertons sur la situation du personnel et notamment aspects triste et des inspecteurs qui rencontre une crise de perte de sens, doublée d'un manque de reconnaissance de leur direction, face à un capitalisme de plus en plus agressifs, nous avons besoin d'une inspection du travail forte pour faire respecter le travail ainsi que celles et ceux qui travaillent, les crédits de fonctionnement pour les services déconcentrés de l'État et donc de l'inspection du travail n'augmente que de 2 % en 2023 si l'effort ne s'accentue pas il y a peu de chances que ces difficultés se résorbent le gouvernement réfléchit-t-il à de nouvelles évolutions de l'organisation de l'inspection du travail, selon le rapport de notre collègue député Pierre Dharréville entre fin 2017 et mars 2022 le nombre des agents chargés du contrôle des entreprises a diminué de 250 équivalents temps plein sur le terrain, cela se traduit par un fort nombre de postes vacants au sein des sections contrôle le taux de vacance serait en moyenne de 15 % cette situation empêche l'inspection du travail de remplir ses missions en certains endroits du territoire et crée des ruptures d'égalité ce budget pour 2023, censé permettre à la France d'atteindre le plein emploi, mais en réalité, nous allons passer du chômage de masse à la précarité de masse pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera donc contre les crédits de la mission Travail et emploi je vous remercie. Merci, j'ai un collègue, la parole est à monsieur Olivier Henno pour huit minutes pour le groupe centriste.

Madame la présidente de commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, d'abord saluer le travail des rapporteurs qui par leurs propos nous ont exposé les réalités de cette mission, ce qu'elle contient, avec plus de 20 milliards d'euros consacré dans ce PLF 2023 la mission Travail emploi est avec la mission Écologie, celle qui enregistre la plus forte progression par l'apport à la loi de finances de 2022, l'analyse de la mission Travail emploi se fait cette année dans un contexte globalement rassurant, on espère que ça durera, sur la question de l'emploi en France, le pays poursuit son recul continu du chômage dont le taux devrait s'établir, selon les prévisions de l'Institut national de la statistique et des études économiques à 7,4 % en fin d'année, nous saluons les efforts déployés depuis plusieurs années pour parvenir au plein emploi, objectif primordial pour notre société, la tendance croissante des crédits de cette mission Travail, emploi et bienvenue pour mener à bien les réformes qui visent à développer les compétences professionnelles des Français et ira à réduire les inégalités d'accès à l'emploi, alors sur l'apprentissage, comme ça a été dit, il faut saluer la progression quantitative, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils ont été cités, il faut aussi saluer le regard qui a changé l'approche culturelle différente sur l'apprentissage pour les jeunes, leurs familles et les entreprises, certes, nous ne sommes pas encore au niveau de, de l'Allemagne, j'aime à raconter le cas de l'entreprise Bayer, cette grande entreprise chimique qui affiche dans son siège, comme 1er chiffrent première fierté le nombre d'apprentis embauchés chaque année au au dépend même du chiffre d'affaires ou du nombre de de salariés, c'est une culture, c'est le modèle rhénan donc pour résumer sur le plan quantitatif les objectifs en nombre d'apprentis sont atteints, mais il y a un mais l'approche qualitative des contrats d'apprentissage signé nous oblige à constater que bon nombre de contrats concernent des bac plus deux bac plus trois voire master, ils sont même devenus pour quelques étudiants pour beaucoup d'étudiants même un moyen de financer des études trop souvent coûteuses alors est-ce le rôle de l'apprentissage, de financer les études, pourquoi pas, mais il y a un certain nombre de conditions à respecter d'abord la clarté des objectifs, hein, et je pense pas que à l'époque du débat sur avenir professionnel nous ayons eu cette vision, les objectifs ont ont légèrement évolué que cela ne se fasse pas aux dépens des de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais les décrocheurs ou des métiers à faible qualification que les métiers en tension et puis bien évidemment qu'on respecte un équilibre financier, alors ça a été dit, hein, mes chers collègues, à ce sujet, lorsqu'on parcourt votre vous rapport on constate que France compétences doit régulièrement recourir à des emprunts qui soulignent certes une dynamique, mais à quel prix, depuis 2020, ces dépenses de guichet dépasse largement le produit des contributions des des employeurs en 2021, le produit de ces contributions s'élève à 8 8 milliards d'euros, alors que les dépenses en faveur de l'alternance représente 9 3 milliards d'euros à ces dépenses s'ajoutent celles liées au compte personnel de formation, estimée à 2,7 milliards d'euros pour 2021 alors sur ce sujet, je vois Martin lévrier il faudra lutter contre la fraude du CPS, bien évidemment, mais aussi réguler à une régulation et et nécessaire sera-t-elle suffisante pour éviter un déficit significatif en 2023 et puis, bien évidemment, il y a la question de de l'équilibre financier d'avenir professionnel alors bref ce déficit de France compétences pour 2023 pourraient être de l'ordre de 4 milliards d'euros, appelant ainsi à de nouveaux emprunts et à des soutiens complémentaire au budget de l'État, une telle situation n'est pas acceptable pour le financement de l'apprentissage et la formation professionnelle et le retour à moyen terme, bien sûr, mais le plus rapidement possible à l'équilibre financier n'est pas une option, c'est une exigence : le programme 100 de retour à l'emploi, lui, baisse légèrement de l'de 5 % en raison des prévisions de diminution du nombre de bénéficiaires en fin de droits à l'assurance chômage dans celui-ci, nous saluons l'augmentation des crédits du secteur de l'IAE, par l'intermédiaire du FIE les acronymes par sa dynamique et la qualité de ces structures qui ont fait leur preuve, ces dernières années, la politique de l'IAE et l'un des outils les plus pertinents pour remettre des hommes et des femmes en situation durable de travail leur action est indispensable si nous voulons collectivement atteint l'objectif de 7 % de demandeurs d'emploi de longue durée, pour ce faire, l'Intelligence des parcours et des accompagnement socio-professionnels doivent être mobilisées afin d'aller chercher celles et ceux qui souffrent de frein à l'emploi et qui en sont les plus éloignés, le programme 102 voix aussi également là. Traduction budgétaire du CEJ créée par la dernière loi de finances, l'accompagnement des quelque 300000 jeunes pour l'année 2023 dont 200000 Bini le nouveau bénéficiaire justifie les quelque 800 millions d'euros prévus. Pour les missions locales et et et celle de Pôle emploi, un mot sur les maisons de l'emploi, ce dispositif, créé par Jean lui pour eau il doit mériter toute notre attention, c'est pourquoi avec Françoise Férat, notre groupe a déposé un amendement pour sécuriser les crédits et les augmenter sur le dispositif territoire zéro, chômeur il fait consensus, le temps de l'expérimentation sera bientôt passer les résultats obtenus sont positifs et conséquent et la limite fixée des 50 communes au territoire est bientôt atteinte et il est temps maintenant de de réfléchir et de décider, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, ce que nous allons faire par rapport aux 134 nouveaux postulants je ne reviens pas sur la question de la future en chômage je crois que le Sénat a bien travaillé sur cette réforme que nous avons eu un bon débat parlementaire, celui d'ailleurs la présence des des 2 ministres pour notre débat sur cette mission, j'ai l'impression que, entre vous, c'est du sérieux, hein, vous êtes présents l'un et l'autre, nous avons bien travaillé sur ces incitations à l'emploi sur la gouvernance sur la VAE aussi, hein, je, je, je, j'insiste sur la vigilance que nous aurons par rapport aux moyens la la VAE qui doit devenir une 3ème voie mais une petite que la formation initiale, la formation continue, le financement du GIP, la question des des sur la gouvernance je réaffirme notre cap, c'est le paritarisme et et le dialogue social et c'est sur ce principe que doit se construire France travaille c'est sur ce principe que nous devons réformer je pense France compétences le déficit de France compétences démontre qu'en matière de bonne gestion, l'étatisation n'est pas une assurance de bonne gestion, bien au contraire, l'étatisation n'est pas la solution et la libéralisation, non plus, il y a une 3ème voie celle du paritarisme et c'est notre cap pour France travaille, mais aussi la réforme de France compétences l'assurance chômage, les retraites Agirc-Arrco le 1 % logement et donc France travail sera regardé comme un symbole de ce point de vue là un dernier mot sur l'inspection du travail, elle est en crise et pourtant dans le monde où l'entreprenariat et parfois un abus, nous avons besoin d'une inspection du travail, forte et l'augmentation de 2 % des crédits avec l'inflation que nous connaissons, paraît bien faible mes chers collègues, pour conclure, je veux dire notre attachement à un service public de l'emploi performant avec une approche personnalisée, le retour à l'emploi des personnes et la éloigné depuis trop longtemps de l'emploi, avec tous les métiers qui sont en tension, le lit chaque jour dans la presse et puis quand on rencontre des des professionnels, hé bien éteinte, un des grands défis de notre pays pour notre pays et c'est pourquoi nous voterons cette mission je vous remercie. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE et pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame, messieurs les Ministres, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier les rapporteurs et et a salué la qu'à la qualité du travail du rapporteur pour avis de notre collègue, Frédérique Puissat, parce qu'il n'est pas forcément aisé d'évaluer la pertinence d'une enveloppe budgétaire dans un contexte d'inflation persistante et des défis considérables pour le travail et l'emploi, il faut donc prendre en compte, dont nos analyses ses nombreuses inconnues pour l'année 2023, protéger les Français, et aller vers le plein emploi, telles sont les ambitions du gouvernement pour 2023, avec une hausse de 6,7 milliards d'euros par rapport à 2022, on note un réel effort pour dynamiser l'embauche des apprentis, il faut donc poursuivre ses efforts déployés depuis 2017 pour parvenir au plein emploi, on est fait, je reste persuadé que le travail est un levier d'insertion incontournable dans notre société, je tiens à saluer, évidemment, les associations, les entreprises et les ateliers d'insertion qui oeuvre au quotidien pour que chacun puisse s'insérer et s'épanouir dans notre société on se sont sont ne peut que se réjouir de la progression des crédits de cette mission, cette tendance haussière reste indispensable pour mener à bien les réformes visant à réduire les inégalités d'accès à l'emploi et à développer les compétences professionnelles de tous les Français. une hausse du budget de la mission Travail emploi doit tout de même être relativisée car il faut prendre en compte dans notre analyse la disparition du programme cohésion de la mission, plan de relance, reviens plus précisément au Crédit du programme sont 2 accès, retour à l'emploi qui sont en légère baisse, soit 5 % en raison des prévisions de diminution du nombre de bénéficiaires des allocations de solidarité des personnes en fin de droits à l'assurance chômage au sein du même programme, il faut souligner l'augmentation des crédits du secteur de l'IAE, par l'intermédiaire du fonds d'inclusion pour l'oncle dans l'emploi, ce qui est en soi une très bonne chose, quelques mots sur la traduction budgétaire du CEJ créée par la dernière loi de finances, les 800 millions d'euros crédits prévus ne devront donc permettre aux missions locales et à Pôle emploi d'accompagner environ 300000 jeunes pour l'année 2023 dont 200000 nouveaux bénéficiaires, ce dispositif hérité du plan de relance doit continuer de monter en puissance afin de permettre. Aux jeunes les plus en difficulté d'entrée de manière pérenne sur le marché du travail, je note aussi une augmentation de 30 millions d'euros pour l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi, ce qui est encouragé, bien évidemment, mais je considère que les crédits consacrés aux entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap reste encore insuffisant. Je poursuis avec les crédits de programme 103 accompagnement pour les des mutations économiques et développement de l'emploi, qui vise à soutenir les actifs et les entreprises dans leur phase de transition et de monter en compétences, on note que les crédits de paiement de ce programme s'élève à 12,6 milliards d'euros, contre 6 milliards dans la loi de finances initiale 2022, la principale hausse concerne évidemment bien évidemment le soutien au développement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, cette hausse des crédits s'explique naturellement par le rapatriement des crédits dédiés à l'activité partielle qui figurait auparavant, dont la mission, plan de relance. Enfin concernant France travaille, je m'interroge sur la pertinence de cette structure car les crédits que nous sommes amenés à analyser vont-ils réellement rééquilibrer les comptes Madame Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle est la situation et quels ajustements sont envisagées pour parvenir à l'équilibre budgétaire, par ailleurs, la question de la gouvernance de France compétences et toujours épineuse qu'on est-il à ce stade, dans l'attente de ces réponses, vous l'aurez compris, tout en restant vigilant le groupe RDSE voteront en grande majorité les crédits de cette mission. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à madame Céline Boutboul ferronnier pour les républicains et pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission Travail et emploi sont examinées dans un contexte bien particulier, où il nous faut respecter un savant jeu d'équilibriste entre la maîtrise des dépenses, d'une part et l'indispensable soutien aux politiques d'emploi, de l'autre le présent budget accompagne situation dans l'emploi globalement favorable, la France connaissant un recul du taux de chômage à 7,4 % actuellement. Cependant, nous sommes toujours mal classés au sein de l'Union européenne, surtout la croissance ne pourra que reculer en 2023 sous les effets conjugués de l'inflation et des problèmes énergétiques, ce qui devrait se répercuter sur le marché du travail, la promesse présidentielle de parvenir au plein emploi, c'est ce quinquennat semble donc malheureusement assez illusoire, comme l'ont souligné d'rapporteur les crédits de la mission évolue à la hausse, mais celle-ci est à relativiser car elle s'explique surtout par la réintégration dans son périmètre de dispositifs porté en 2021 et 2022 par le plan de relance notamment les aides à l'apprentissage et l'activité partielle, en tenant compte des loi rectificative votée en 2022, les Budgets de cette année de l'année prochaine serait même très proche, contrairement aux messages diffusés par le gouvernement concernant les réformes envisagées, je voudrais formulé plusieurs réserves et interrogations, monsieur le Ministre, vous avez annoncé une réforme du service public de l'emploi, avec la création d'un nouvel organisme France travaille, il s'agit de simplifier les parcours en mettant en commun les informations et stratégie d'accompagnement, notamment avec un point d'entrée unique dans le service public de l'emploi, les différents acteurs auditionnés au Sénat ont exprimé leurs réserves, estimant le projet de loi très flou, il ne dispose d'aucun élément précis sur son périmètre et son contenu une concertation a été engagée, mais elle manque de transparence dans ses objectifs et elle n'associe pas le Parlement, nous serons donc extrêmement vigilants pour éviter que cette nouvelle structure ne se transforme en usine à gaz ou ne soumettre les différents opérateurs à des contraintes inappropriée, vous avez dans lancé par ailleurs une expérimentation concernant les bénéficiaires du RSA qui dépend précisément de la création de France travaille, l'organisme sera chargé de mettre en place un contrôle et un accompagnement renforcé, nous sommes favorables à un suivi qui soit enfin efficace, la Cour des comptes vient en effet de pointer les défaillances du dispositif d'accompagnement en matière de retour à l'emploi, la moitié des allocataires du RSA le sont encore, au bout de 4 ans et 29 % après 7 ans, un budget de 20 millions d'euros, est prévue pour le lancement de l'expérimentation dans une dizaine de territoires pilotes sur 12 mois, on peut se demander si l'expérimentation puis sa généralisation pourront se conduire à moyens constants sur le terrain, à l'image de nos rapporteurs je souhaiterais faire part de notre inquiétude concernant France compétences, structure créée en 2018 pour réformer la formation professionnelle France compétences a bénéficier de transferts de trésorerie exceptionnelle dans les de loi de finances rectificative de cette année, malgré cet apport s'élevant à 4 milliards d'euros, son déficit pourrait atteindre 3 4 milliards d'euros en 2022, la Cour des comptes s'alarme d'une impasse financière, selon ses propres termes, le déficit est clairement lié à la réforme du financement de l'apprentissage sous le précédent quinquennat depuis 2020 les CFA sont financés par les entreprises en fonction du nombre de contrats signés et l'État s'est substitué aux régions pour compléter ce financement la poule type éducation des contrats d'apprentissage fait basculer France compétences dans le rouge. Les crédits que nous sommes une nouvelle fois invité à voter pour rééquilibrer ses comptes interroges sur le fonctionnement et la pertinence de la structure notre groupe soutiendra donc l'amendement de la rapporteure de la commission des affaires sociales, Frédérique Puissat, dont nous saluons la qualité du travail et qui vise à réguler les dépenses de France compétences de même nous suivrons son avis éclairé pour dégager des économies sur les des crédits affectés au pic, celui-ci n'ayant pas démontré son utilité en matière d'insertion et de formation professionnelle et devant prendre fin l'année prochaine l'économie totale réalisé seraient ainsi de 800 millions d'euros, ces mesures sont pleinement cohérente avec notre préoccupation de maîtrise des dépenses publiques de l'État, je souhaiterais enfin évoquer la relance de l'apprentissage, je me réjouis que la dynamique se poursuivent avec une hausse de 38 % du nombre de contrats entre 2020 et 2021, le gouvernement prévoit la signature de plus de 800000 contrats cette année, contribuant à améliorer l'emploi des jeunes, ce succès est en partie due aux aides qui ont été versées dans le cadre de la crise sanitaire, je m'interroge donc sur l'éventuelle suppression le 31 décembre prochain de l'aide à l'embauche d'apprentis de plus de 18 ans. Cette aide exceptionnelle contribue à relancer l'attractivité de nombreux métiers, je pense notamment à la filière agricole 40 % des agriculteurs ont plus de 55 ans et partiront à la retraite d'ici à 2030 alors que seul un départ sur 3 et remplacer les petites structures agricoles ne pourront plus recruter d'apprentis sans cette aide à l'embauche qui couvre la première année de salaire, je tenais à rappeler cette situation à la veille de concertation menée avec les partenaires sociaux et souhaiterait avoir votre sentiment sur ce point, monsieur le Ministre, le groupe Les Républicains votera ce budget en augmentation, avec les mesures d'économies que nous avons indiqué notre groupe souhaite que l'examen de la loi de finances permette de faire bouger les lignes tracées par le gouvernement, nous visons ainsi un budget maîtrisé, tenant compte des difficultés actuelles mais protégeant notre pays d'une dette devenant abyssal : protéger les Français et leurs employes passe aussi et surtout par cette discipline, je vous remercie. La parole est maintenant à Joël Guerriau pour le groupe des indépendants et pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à tendre le plein emploi, c'est à la fois un objectif économique et social, économique, évidemment, car davantage d'emplois, c'est un accroissement d'activité s'accompagnant d'une meilleure intégration par le travail social aussi parce qu'un accroissement d'activité, c'est davantage de recettes publiques pour financer la solidarité, ce sont les entreprises qui nous permettront d'atteindre cet objectif, et je l'espère d'ici la fin du quinquennat il n'y a pas d'emplois durables, que la création de valeur ajoutée, c'est d'abord sur les entrepreneurs et les travailleurs que nous comptons pour y parvenir, mais la puissance publique peut et doit aider à atteindre le plein emploi, notamment en facilitant l'intégration des publics les plus éloignés du marché du travail ces leviers d'action se trouve dans la mission que nous examinons, aujourd'hui, les crédits de la mission Travail emploi dépasse cette année les 20 milliards d'euros, ils augmentent de près de 29 % par rapport à la loi de finances initiale et c'est bien sûr considérable mais cette hausse appelle plusieurs remarques : la première, c'est l'effort de sincérité budgétaire du gouvernement, en effet, les crédits inscrits dans cette mission pour 2023 sont largement supérieurs à ceux inscrits à la loi de finances initiale pour 2022, mais pour autant, ils sont nettement inférieurs à ceux, finalement débloqué en 2022 après les 2 projets de loi de finances rectificative c'est pourquoi si et seulement si, en cours d'année, les crédits de la mission ne sont pas significativement augmenté par la voie d'un projet de loi de finances rectificative alors le gouvernement aura finalement maîtrisé la dépense associé la 2ème remarque répond à des interrogations exprimées par plusieurs de nos collègues, en effet, alors que la vocation des politiques budgété dans cette mission est de stimuler l'emploi, on pourrait penser que les crédits sont amenés à diminuer lorsque la situation du marché du travail s'améliore, mais la situation n'est pas si évidente, et pour cause, la plupart des mécanismes déployés par le gouvernement pour faciliter l'intégration par le travail sont plus structurels que conjoncturels, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à se maintenir, sans tenir compte de la situation du marché de l'emploi, cela m'amène à ma 3ème et dernière remarque qui concerne l'apprentissage nous sommes nombreux ici à soutenir depuis longtemps l'apprentissage comme vecteur d'intégration des jeunes au marché du travail, le gouvernement a mis les bouchées doubles pour encourager les entreprises à embaucher des jeunes, et les résultats sont nets : le nombre d'entrées en apprentissage, a doublé entre 2000 19 et 2021 passant de 370000 à 740000 jeunes le montant des aides à l'embauche de alternant est ainsi passé de 1,3 milliards d'euros en 2020 à 4 5 milliards en 2021 sur ce point, je partage, analyse de notre rapporteur spécial Emmanuel Capus, dont je tiens à saluer le travail, il faut à la fois reconnaître le succès de l'apprentissage et poser la question de l'efficacité de la dépense publique, le gouvernement a engagé avec les partenaires sociaux, des négociations sur ce sujet et cette dynamique de dialogues me semble positive, je l'ai dit d'emblée le seul emploi durable, c'est la création de valeur ajoutée pour les entreprises, l'emploi aidé améliore les statistiques du chômage mais elle pèse sur les finances publiques et masque la compétitivité réelle du pays, l'apprentissage ne doit donc pas être une nouvelle forme d'emplois aidés, avec des effets d'aubaine aussi pour les entreprises. Cependant Monsieur le Ministre, j'espère que Bercy ne cédera pas à la tentation d'une approche strictement budgétaires pour évaluer le dispositif de l'apprentissage, beaucoup d'effets positifs, notamment au plan de la cohésion sociale et de l'éducation des jeunes n'apparaîtront jamais dans les comptes mais sont extrêmement précieux, je souhaiterais enfin ajouter un mot sur les mécanismes de soutien aux entreprises adaptées, contrairement au dispositif financé par la mission qui permettent l'intégration par le travail et doivent répondre aux logiques du marché ces crédits répondent d'un impératif éthique, permettre aux personnes en situation de handicap de trouver leur place dans la société d'contribuer par leur travail, de se sentir utile au quotidien, tout cela rend notre société plus humaine et plus équitable, c'est pourquoi je tiens à saluer l'augmentation des dotations en faveur de l'emploi des personnes handicapées à hauteur de 467 millions d'euros, soit une progression de près de 9 % par rapport à 2022 ces aides seront complétés comme l'an dernier par une contribution de l'Agefip de 50 millions d'euros, notre groupe votera les crédits de cette mission, sous réserve de l'adoption des amendements proposés par nos rapporteurs spéciaux, merci de votre attention. Merci, la parole était ensuite Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe Écologie Solidarité territoire dans cinq minutes.

Monsieur le président, monsieur le Ministre, chers collègues, quelques semaines seulement après que le gouvernement est officialisé la contre-réforme de l'assurance chômage, nous nous trouvons face à un texte qui amorce sa mise en oeuvre ainsi 20 millions d'euros sont alloués à l'expérimentation France travail dont les contours et l'émission reste flou, si ce n'est de répondre à l'injonction du travailler plus et qui se met progressivement en place, sans que ni le parlement ni les partenaires sociaux ne soient pleinement saisi du contenu du projet ce 49 3 de l'expérimentation. Vice-peut être à nous mettent nous et les partenaires. Sociaux devant le fait accompli lorsque la convention tripartite Pôle emploi État Unédic dont la reconduction est en train de discuter prendra définitivement fin, elle se terminera d'ailleurs sans que le gouvernement n'a été à la hauteur de ses promesses budgétaires, soit lors de la signature de la convention en 2015 de 1 virgule 5 milliards d'euros, alors que le financement est aujourd'hui de 1,2 milliards et la hausse des crédits alloués cette année à Pôle emploi n'est qu'un rattrapage d'année consécutive d'austérité de baisse des effectifs, l'État transfère un peu à peu la charge du pôle emploi sur l'Unédic, donc au détriment des prestations qu'il convient alors de diminuer la pérennisation des ETP accordée à Pôle Emploi pour la mise en oeuvre du contrat d'engagement jeune en 2020 et qui explique la hausse actuelle des crédits doit améliorer la dégradation constante des conditions de travail au sein de l'Agence souci. Les écologistes se poseront à leur réduction car, selon les syndicats, la proportion de personnels en CDD à Pôle emploi serait passé de 5 % environ en 2019 à 13 % en 2021, avec de fortes disparités locales puisque certains sites peuvent atteindre jusqu'à 50 chargé de l'emploi en France diffuse le CDD comme norme aussi en 2017 chaque conseiller avait en moyenne en portefeuille 46 demandeurs d'emploi en accompagnement global aujourd'hui 54 et 336 en accompagnement suivi aujourd'hui 406, de l'avis général, les réformes successives ont porté atteinte à la sécurité des agents provoquer des pertes de sens au travail et une gestion parfois erratique des dossiers du fait de changements incessants de calcul des indemnités. le gouvernement se réjouit de la baisse du chômage en partie en trompe oeil et baisse en conséquence, les crédits du programme 102 accèdent accès et retour à l'emploi, or de l'avis même de un tiers de la hausse du taux d'activité mi-2022 résulte des contrats en alternance, notamment en apprentissage, soit des emplois hautement subventionnés profitant largement, selon la Cour des comptes aux plus diplômés et non et non au 1 virgule 5 millions de jeunes sans emploi ni formation ces derniers dépendent en réalité des contrats emplois-jeunes qui, malgré un certain succès avec près de 200000 contrats en 2022 reste en nombre insuffisant en projection 2023 et comme toutes personnes éloignées de l'emploi, ils dépendent beaucoup des emplois aidés comme les parcours emploi Compétences qui eux sont en diminution de 20000 passe de 12 à 6 mois, réduisant ainsi leur durée totale maximale à dix-huit mois cela sans explication ni justification. De plus, la baisse du chômage pour 2023 est une hypothèse assez hasardeuse qui ne tient pas compte des travaux de l'Unédic, prévoyant un tassement de la progression des emplois salariés dès l'année prochaine comme de lait l'OFCE qui tablent sur une remontée du chômage jusqu'en 2000 vingt-quatre dans le contexte où la réforme de l'assurance chômage aura pour effet de rendre les fins de droits, plus précoce et de réaliser plusieurs milliards d'économies, la mission certes présente des crédits en hausse, mais peut être faussement car la hausse de la mission 103 par exemple et du très largement transfère des crédits dédiés à l'activité partielle qui figurait auparavant dans la mission, plan de relance, passant de 11 9 milliards contre 7 au PLF 2023. Ceci pour les autorisations d'engagement et pareil pour les crédits de paiement ces jeux budgétaire ne masque pas les insuffisances d'une politique de l'emploi qui reste antisocial tournés vers vers la baisse des droits des demandeurs d'emploi en conséquence le groupe écologiste solidarité et territoires ne votera pas les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci, cher collègue, il a parole est maintenant à Martin lévrier pour le groupe RDPI. Et pour six minutes. Bien.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, le plein emploi n'est pas une utopie, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail a baissé de 2 2, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron pour atteindre son niveau le plus bas depuis 15 ans le gouvernement porte l'ambition du plein emploi et les crédits dont la mission Travail, emploi et doté le démontre, ils atteignent un montant total de 20,29 milliards d'euros en autorisations d'engagement, soit une hausse de 28 % et de 20,88 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 42,57 %. Cette hausse de près de 6,2 milliards d'euros en crédits de paiement s'explique marge majoritairement par des changements de périmètres des dispositions jusque là financés par le plan de relance, à l'instar de la prime à l'apprentissage et d'une partie de l'activité partielle, font désormais l'objet d'un financement de droit commun, notons qu'à périmètre comparable, l'augmentation est de 1,1 milliard d'euros en crédits de paiement est d'environ un milliard d'euros en autorisations d'engagement du à la dynamique de compensation des exonérations de cotisations qui représente, pardon, un peu plus de 6 1000000 600 millions d'euros par les emplois créés en 2022 l'inscription de 350 millions d'euros au titre de la partie formation du Front national pour l'emploi et 50 millions d'euros pour les financements de dispositifs de transition collective. Afin de bien mesurer la portée de ces crédits, les moyens les plus efficaces et, dans le lycée, les principes dans listés par dans les principales modifications par rapport à l'année précédente, notons le renforcement de la prévention en santé au travail suite à la mise en oeuvre de la loi du 2 août 2021, je le disais juste avant l'inscription en droit commun de 350 millions d'euros au titre du FNE, formation et des dispositifs de transition collective jusque-là financées dans le cadre du plan de relance la poursuite du financement du programme d'investissement dans les compétences de 5 milliards d'euros, dont un virgule 6 milliards d'euros pour financer le vote régional, l'augmentation du budget de l'insertion par l'activité économique afin de financer une augmentation de 702 7000 ETP en structures d'insertion, l'objectif du gouvernement étant d'atteindre 240000 bénéficiaires, le renouvellement des crédits pour l'accès des jeunes à l'emploi, avec l'objectif de 300000 contrats d'engagement jeune une aide aux missions locales, avec un budget de plus de 630 millions d'euros, mes chers collègues, le travail mené à bien par les gouvernements qui se sont succédé depuis 5 ans, porte ses fruits, nous devons donc continuer selon les mêmes principes et non chercher à Rabat a raboté arbitrairement certaines dépenses combattre le chômage, pour atteindre le plein emploi n'est pas une charge, c'est un investissement, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons accepter le premier amendement de Madame la rapporteure qui réduit les crédits à hauteur de 850 millions d'euros en autorisations d'engagement et 600 millions pendant huit cents quant au second il et une proposition d'un rapport France compétences face à une crise de croissance, il en détourne en partie le sens si l'idée d'un reste à charge pour certaines formations a été évoqué cette afin que les partenaires sociaux s'en emparent et propose des solutions permis cette démarche nous paraissait plus cohérente, même si cet amendement va dans la bonne direction, mes chers collègues, je le redis dans ce nouveau contexte qui casse les habitudes de la gestion du chômage de masse, nous devons continuer à investir dans toutes les solutions pertinentes pour atteindre le plein emploi, avant de conclure : je rappellerai Les 8 chantiers identifiés comme prioritaires par le ministère au cours des prochaines années et pour lesquels il nous faudra travailler en bonne Intelligence, la rénovation du service public de l'emploi par la création de France de la réforme de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et la meilleure insertion des publics les plus éloignés de l'emploi, la poursuite du déploiement du contrat d'engagement jeune le perfectionnement de l'assurance chômage, l'amplification de la dynamique de l'apprentissage, la préparation des actifs aux compétences de demain et bien entendu le soutien de l'emploi des seniors et la garantie de l'avenir de notre système de retraite. Mes chers collègues pour parvenir au plein, en plein emploi, l'État est pleinement mobilisé, bien que très attentif à la maîtrise des dépenses publiques, il donne au travers de ses Budgets de solides garanties et des moyens sans précédent pour que chacun puisse accéder à l'emploi ou s'y maintenir, et que chaque entreprise et les compétences nécessaires aux métiers de demain c'est donc bien naturellement que le groupe RDPI votera les crédits de la mission. Merci, cher collègue, et la parole enfin État monsieur Édouard Courtial pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances Madame messieurs les rapporteurs, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, le travail plutôt que l'assistanat, le sens de l'effort plutôt que le nivellement par le bas, le mérite, l'équilibre des droits et les devoirs, voilà les valeurs que notre groupe porte et assume dans cet hémicycle et sur le terrain, cela se traduit par les propositions que nous faisons sur cette mission et l'analyse que nous en tirons les crédits qui je le rappelle, finance principalement des dispositifs concourant à la politique de l'emploi et qui enregistre une très forte augmentation, ils s'inscrivent dans un contexte particulièrement favorable qui doit être indéniablement, lui, en effet, la situation de l'emploi s'est amélioré par rapport à fin 2019, l'emploi salarié a progressé 800000 personnes et le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de près de 400000 la dépense budgétaire, porté par la mission s'est alourdi, mais d'autres dépenses ont diminué, notamment l'indemnisation du chômage, l'Unédic sera en excédent cette année pour la première fois depuis 2008, quant à la progression de la masse salariale, elle se répercute évidemment sur les recettes de l'État et des organismes de protection sociale en outre les des moyens très importants ont été consacrés ces 3 ou 4 dernières années à des dispositifs dont beaucoup étaient antérieurs à la crise, d'autres mises en place durant la crise mais destiné à être en partie pérennisée, notamment en direction des jeunes ou des chômeurs de longue durée, ainsi les moyens qui leur sont alloués progresse de plus de 15 % il est à noter la montée en charge du contrat engagement jeune avec un objectif de 300000 pour 2023 les premières données sur le déploiement des CEJ sont d'ailleurs encourageantes, s'il est encore trop tôt pour mesurer son effet sur l'insertion professionnelle des jeunes, les objectifs fixés paraisse cohérent et exigeront d'assurer la bonne articulation des CEJ avec les autres dispositifs d'insertion des jeunes, en particulier dans le cadre du projet France travail dont l'objectif est d'harmoniser les les actions d'accompagnement vers l'emploi, l'inclusion des personnes en situation de handicap par le travail est une absolue nécessité, comme la commission, j'appelle à l'adoption de l'Arctique permettant de prolonger les expérimentations favorisant l'emploi de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées partagent également les réserves de rapporteur quand le quant à l'opportunité de maintenir les emplois francs dont les premières évaluations n'ont pas permis de mesurer l'impact sur l'emploi dans les QPV, mais je suis particulièrement favorable à la hausse des compensation des exonérations de cotisations sociales sur les entreprises, particulièrement en faveur des services d'aide à domicile et la déduction des heures supplémentaires, dispositif Tepa dont les républicains sont à l'origine, les enjeux sur ces 2 points pour nos compatriotes sont majeurs, le 1er dans un contexte de vieillissement de la population et le second dans le contexte économique que nous connaissons, enfin, je tiens à me féliciter du succès de l'apprentissage qui est essentiel, malgré le poids financier qui représente, il enregistre une véritable dynamique positive avec une hausse de 38 % des contrats entre 2020 et 2021, c'est un atout pour notre jeunesse et un dispositif plébiscité par nos entreprises, surtout dans nos territoires ruraux, néanmoins, il est indéniable qu'il nous faut réfléchir la soutenabilité du financement qui représente un enjeu majeur, il repose sur la prise en charge des contrats selon un niveau déterminé par les branches professionnelles est assurée par France compétences dont les ressources sont principalement issus des contributions des employeurs à la formation professionnelle et à l'apprentissage, or depuis 2020, ces dépenses de guichets dépasse largement le produit des contributions des employeurs et face à ce déséquilibre chronique France compétences doit régulièrement recourir à des emprunts de court terme pour faire face à ses besoins de trésorerie ainsi le PLF pour 2023 demandent une enveloppe de 1,68 milliards d'euros pour l'établissement, à cette dotation s'ajoute un ensemble de mesures qui permettraient de limiter les dépenses de l'opérateur pour conclure, permettez-moi 2 observations : la première concerne le CPF, dont la visibilité et l'effectivité doivent être améliorées, des mesures de régulation de l'offre des formations éligibles fort justement été engagée par le contrôle des certifications professionnelles, la lutte contre la fraude au CPF qui serait renforcée par une proposition de loi en cours de discussion constituerait un levier supplémentaire dont les effets sont toutefois difficile à évaluer, en outre, l'article 49 du PLF introduit à l'Assemblée nationale, propose que la mobilisation du CPF par son titulaire pour le financement d'une action de formation fassent l'objet d'un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret, il est souhaitable de réguler les dépensiers au CPF afin de recentrer le dispositif sur l'employabilité des utilisateurs et sur le développement des compétences à finalité professionnelle, je suis donc favorable à l'amendement adopté instaurant un plafonnement de la prise en charge du coût de certaines formations pour recentrer et rendent plus efficace le dispositif, je défends aussi dans une proposition de loi déposée que signée par de nombreux collègues de mieux lutter contre le démarchage téléphonique abusif qui touche spécialement le CPF la seconde, et de rappeler que l'argent public, ce n'est pas de l'argent gratuit mais le fruit du travail des Français du bon sens, me direz-vous, et vous aurez raison ce qui justifie d'ailleurs l'amendement notre collègue Frédérique Puissat ainsi, dans le contexte économique et financier actuel, cela oblige l'état, en particulier à faire preuve d'exemplarité et d'efficacité dans l'engagement des dépenses, à ce titre, il serait sage, qu'il s'applique à lui-même les efforts qu'il exige des collectivités locales mieux faire avec moins, est devenu, année après année le leitmotiv forcer les collectivités que les élus sur le terrain en première ligne, applique avec détermination et courage, je vous remercie. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à monsieur Olivier Dussopt Ministre du Travail du plein emploi, de l'insertion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Carole mais, mais Madame et messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le président, la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, le professeur de budget que nous vous présentons avec Carole Granjean augmente, comme cela a été dit, de 4 virgule 5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 6,2 milliards d'euros en crédits de paiement entre le budget initial pour 2 1000 22 et le budget initial pour 2023, mais cela a été dit aussi en 1er par le rapporteur, cette évolution est peu significatif pour 2 raisons : plusieurs dispositifs étaient financés sur l'urgence et sur la relance, comme les aides à l'apprentissage que nous maintenons et la mission Travail et emploi à bénéficier de plus de 7 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2007 milliards d'euros en crédits de paiement à l'occasion de la loi de finances rectificative du mois de juin dernier, au total, le budget du ministère bénéficiera donc de 20 viril 3 milliards d'euros en autorisations d'engagement de 20 virgule 9 milliards d'euros en crédits de paiement et avec un seul objectif : derrière ce chiffre, la poursuite du plein emploi et l'atteinte du plein emploi, ce budget est un budget de plein emploi, d'abord parce qu'il traduit les effets de la baisse du chômage ainsi les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique financée par l'État, ce sont 80000 de moins que ce que nous redoutions l'année dernière, ce qui nous permet d'économiser 492 millions d'euros, ce qui se traduit aussi par une baisse des crédits cette action, nouvelle, bonne nouvelle parce que cette baisse du nombre d'allocataires n'a pas, n'a pas été accompagnée d'une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, c'est donc du retour à l'emploi et ainsi 156000 demandeurs d'emploi de très longue durée ont retrouvé le chemin de l'emploi au cours de la dernière année, c'est aussi un budget de plein emploi, parce qu'il encourage l'emploi des jeunes ainsi l'alternance mais Carole Grandjean il reviendra voit ses crédits augmenter de 3,5 milliards d'euros consacrés à l'aide à l'embauche d'alternance, c'est pour cette raison et parce que nous connaissons cette dynamique en matière d'apprentissage et d'alternance que le président de la République et le gouvernement se sont fixé un objectif d'un 1000000 d'apprentis en 2027, c'est ce qui explique la mobilisation du gouvernement des services des opérateurs de l'emploi, certains considèrent que l'emboutissage coûte très cher, nous, nous pensons que le plein emploi, rapporte et que l'apprentissage est un levier majeur pour atteindre cet objectif de la même manière, le budget initial de l'État soutient pour la première fois la trésorerie de France compétences par l'octroi d'une subvention de 1,7 milliards d'euros, le soutien est même supérieur à 2 milliards d'euros, lorsque l'on intègre la prise en charge par l'état du versement aux régions des crédits nécessaires au financement des pactes régionaux dans le cadre du pic, je veux saluer les efforts, la volonté de régulation, même si nous ne partageons pas la méthode consistant à diminuer des crédits, tels que la commission des affaires sociales, le propose et je veux saluer le rapport sénatorial dont Madame la rapporteure, est une des auteurs pour nous aider, nous accompagner sur le chemin du rétablissement des comptes de France compétences ce budget encourage aussi le plein emploi, parce qu'il favorise les compétences pour développer l'emploi, d'aujourd'hui et l'emploi de demain, nous prévoyons dans ce budget 300 millions d'euros du FN information 50 millions d'euros, dispositif de transition collectif car nous sommes con, convaincu qu'il faut former pour réduire les tensions actuellement visible sur le marché du travail en matière de recrutement, mais aussi pour développer les compétences indispensables pour accompagner les transitions de fond de notre économie dans le secteur de la santé, mais je pense bien évidemment aux transition énergétique ou numérique, je veux aussi souligner que ce budget et le budget de l'emploi pour tous et en particulier le budget de celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, c'est la raison pour laquelle 2023 sera une année de transition marquée par l'installation progressive de France travaille, vous avez été nombreux à souligner votre curiosité, votre impatience de connaître la maquette, le détail de la création de France travaille sans répéter ce que j'ai déjà dit, le fait que ce ne sera pas une opération de fusion ou de rapprochement, de structures, nous ne voulons pas connaître l'embolie l'embolie connaît connu au moment de la création de de Pôle emploi, il a maintenant plus de 10 ans, mais cette maquette et ces détails seront présentées à l'occasion de la fin de la préfiguration que nous avons confié à Thibault guili en la fin du mois de décembre et et le milieu du mois de janvier, dans ce contexte nous avons préservé les moyens de Pôle emploi alors même que le chômage a diminué et, ainsi, en 2023 nous accordera une subvention d'1,250 1000000, 1,250 milliard d'euros à Pôle emploi niveau subventions qui n'avait pas athée atteint depuis 2019, cela permet de pérenniser les effectifs accordée à l'opérateur pour la mise en oeuvre du contrat engagement jeune, cela permet de poursuivent le déploiement du parcours de remobilisation des demandeurs d'emplois et le maintien de la mobilisation au service des entreprises dans un contexte de fortes tensions de recrutement, c'est la raison pour laquelle les effectifs de Pôle Emploi resteront stables, avec une baisse limitée à 31 DTP, sur un total de 48850 voire 52900 si l'on prend en compte les emplois hors plafond pour l'essentiel des CDD ainsi Pôle emploi est armés pour la bataille du plein emploi en 2017, les recettes de Pôle Emploi s'est levé à 5 3 milliards d'euros or pactes régionaux et ses actifs, ses effectifs à 49918 personnes en 2000 en 2023 les ressources de Pôle Emploi seront de Cyril 5 milliards d'euros et ses effectifs globaux de 52840 TP pourquoi est-ce que nous maintenons ces ces moyens pourquoi est-ce que nous augmentons la subvention en faveur de de Pôle emploi parce que nous croyons au renforcement de l'accompagnement pour le pour le pour le plein emploi, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons aussi préserver, par ailleurs, les crédits de lutte contre la pauvreté ou des crédits accompagnant les expérimentations de service public de l'insertion et de l'emploi avec, en 2023 29 millions d'euros en autorisations d'engagement et 39 ans en crédits de paiement en matière d'accompagnement dans l'emploi des plus éloignés de l'emploi, je veux dire un mot de l'insertion par l'activité économique, d'abord pour rappeler que ces 3 dernières années, le budget de l'IAE a fortement augmenté de plus de 400 millions d'euros dans le cadre du pacte pour l'ambition de l'insertion par l'activité économique 2023 et là aussi une année de consolidation et nous ne nous nous maintenons néanmoins un budget en hausse à hauteur de 1 virgule 3 milliards d'euros, 1 virgule 3 milliards d'euros pour l'insertion par l'activité économique, c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint et qui marquent une augmentation des crédits par rapport à ce qui sera réalisé en 2022 réalisations inférieur à la prévision, puisque même ses structures connaissent des difficultés de recrutement qui peuvent expliquer ce le fait que tous les crédits ne seront pas consommés, cela permettra de financer en 2023, plus de postes que le nombre de postes financés réellement et effectivement en 2022 je veux aussi souligner que le pic a eux pour favoriser la formation des salariés en insertion et lui non seulement prolongé mais augmenté de 25 % en 2023 puisqu'il passe de 80 à 100 millions d'euros, toujours pour aller vers le plein emploi et permettent l'emploi de tous, je tiens à souligner devant vous, le fait que les entreprises adaptées bénéficieront pour ce qui les concerne de plus de 500 millions d'euros dans 15 millions de reconduction du fonds d'accompagnement et de transformation des entreprises adaptées, nous allons aussi en même temps, poursuit les efforts pour les jeunes éloignés du marché du travail et nous reconduisons l'objectif de 300000 bénéficiaires du contrat engagement jeune pour l'année prochaine avec l'accompagnement nécessaire, ce qui signifie un hein 1,76 milliards d'euros qui sont inscrits au au projet de loi de finances pour se faire, enfin, je tiens à rappeler, a souligné que les contrats aidés, reste un outil traditionnellement utilisée dans les politiques de l'emploi en 2023 le nombre de contrats aidés diminuera pour le secteur marchand et c'est un point que nous assumons le marché du travail va mieux et d'autres dispositifs de soutien à l'emploi se développe par ailleurs hein si nous prévoyons 31100 100 150 CIE pour 2023 contre 53200 en 2022, par contre, nous prévoyons un total de 80000 les contrats des les contrats aidés, pour lui, le secteur public, contre 77700 en 2022, nous savons que ces contrats sont particulièrement utile aux collectivités locales, au delà de ses grandes priorités et de ses grandes lignes d'action, je souhaite aussi souligner que le plein emploi est aussi le bon emploi, c'est la raison pour laquelle le programme 111, améliorer la qualité de l'emploi et des relations du travail sera augmenté de 16 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 18 millions d'euros en crédits de paiement notamment pour accompagner la modernisation des services de prévention de santé au travail, enfin pour mettre en oeuvre ces politiques le ministère peut compter sur des agents dévoué engagée de grande qualité en 2023 pour la première fois depuis plus de 10 ans les effectifs du ministère augmente avec un schéma en hausse de 60 ETP, ce qui permettra de renforcer, d'une part, les services du ministère, notamment anti-du renforcement du pilotage des politiques publiques et la réinternalisation de mission de prestataires externes, cela permettra d'accompagner la préparation des Jeux olympiques et de gérer notamment les demandes de dérogations au droit du travail en matière d'organisation des Jeux et de présence des entreprises prestataires, cela permettra aussi d'accorder des moyens nécessaires au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'État entre 2011 et 2021, le schéma d'emplois était négatif d'environ 180 ITT par an en moyenne, il a été stabilisé en 2022 à 0 je dois cependant souligner pour la clarté des débats que le plafond d'emplois est lui en baisse de 188 équivalents temps plein par rapport à 2022, pour s'établir à 7773 équivalents temps plein, cela s'explique par le maintien obtenu des renforts exceptionnels dans les services des le qui devaient disparaître en 2023 et que nous maintenons pour partie la décrue sera donc progressive, ce qui nous permettra, pour les services du ministère du Travail, de l'absorber plus facilement que si cette ces moyens avait été supprimé en une seule fois, ainsi 105 équivalents temps plein sur les 210 sont conservées aussi de l'accompagnement des restructurations économiques et cent vingt équivalents temps plein sur 160 sont maintenus otite, des mesures de correction en matière de mise en oeuvre de la nouvelle organisation territoriale de l'État j'en reste là pour céder la parole à Carole Grandjean sur les questions de formation et d'apprentissage, je vais simplement pour conclure remercier les 3 rapporteurs spéciaux du Sénat, ainsi que l'ensemble des sénateurs membres des 2 commissions qui ont examiné ces textes pour la qualité de leur travail et je crois la richesse et la sincérité de nos échanges. Merci monsieur le ministre, donc la parole pour les cinq minutes restantes et que Madame Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle. Monsieur le président, Monsieur le, le ministre du Travail du plein emploi et de l'insertion, cher Olivier, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs madame la rapporteure pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, le budget que que nous vous présentons aujourd'hui encourage pleinement l'emploi des jeunes, l'emploi de long terme parce qu'il encourage aussi l'alternance, ce sont 3 5 milliards d'euros qui sont investis en crédits de paiement et de 3 milliards d'euros en autorisations d'engagement qui sont consacrés dans ce budget initial aux aides à l'embauche d'alternants, c'est une somme importante que nous assumons, car c'est un investissement à la fois dans l'éducation des jeunes et dans les compétences des entreprises, le président de la République, effectivement, et le gouvernement sont fixés un objectif d'un 1000000 d'apprentis par an d'ici à 2027 nous sommes pleinement mobilisés vers l'objectif de faire en fin de la France une nation de l'apprentissage à tous les niveaux de qualification et dans toutes les entreprises, il est clair, comme vous l'avez indiqué mesdames et messieurs les rapporteurs que le développement de l'apprentissage, a conduit à une hausse des dépenses et un déséquilibre financier de France compétences dont le financement à l'alternance s'élève à plus de 10 milliards d'euros, je tiens à le dire, nous assumons car les résultats sont sans appel : le taux d'insertion dans l'emploi a fortement contribué à diminuer le taux de chômage des jeunes, sur ce point, l'apprentissage est une réussite, fortes, notamment pour les moins qualifiés d'entre nos jeunes et nous constatons qu'effectivement 72 % des jeunes trouvent un emploi durable, suite à leur apprentissage, nous avons appliqué dès cet été, des mesures de régulation des dépenses en concertation avec les branches professionnelles qui a conduit à un mouvement général mais non uniforme de baisse des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage afin de les rapprocher des coûts observés, l'objectif n'était pas d'appliquer une stricte mesure d'économie, mais bien de ramener les niveaux de financement des contrats au juste prix celui constaté dans les CFA, par le biais de l'analyse de leur comptabilité analytique enfin ensuite les primes exceptionnelles de l'État, décidé dans le contexte de crise sanitaire et qui ont permis de soutenir la formation des jeunes arrivent à échéance à la fin de l'année 2023 et vous l'avez rappelé mesdames et messieurs les sénateurs, et donc des concertations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d'un calibrage plus adapté plus adapté pour la suite, en outre, nous souhaitons soutenir la trésorerie de l'opérateur et pour cela, le gouvernement a octroyé 2 milliards d'euros en PLFR de fin de gestion au bénéfice de France compétences ce montant s'ajoute aux 2 7 milliards d'euros déjà octroyés par l'État en 2021 sur la LFI 2 21 aux 2 milliards d'euros, ouvert en 2022 par le PLFR 2022 de cet été et au 1 virgule 7 milliards d'euros, qui est proposé d'ouvrir en PLF 2023 2000 2 milliards d'euros de soutien avec la rebudgétisation de la moitié des pactes régionaux. Je voudrais mesdames et messieurs les sénateurs, revenir un instant sur le compte personnel de formation la dépense 2022 sera stabilisé par rapport à la dépense 2021 à 2 7 milliards d'euros environ, alors qu'elle avait fortement augmenté en 2020 c'est donc en cohérence avec nos objectifs ambitieux pour la jeunesse et en responsabilité vis à vis de France compétences que l'État agit l'article 49 adopté à l'Assemblée nationale et que Madame et messieurs les rapporteurs, vous avez souhaité préciser par amendement présente un mécanisme de régulation qui vient compléter l'ensemble des mesures déjà mises en place par le gouvernement pour mieux orienter les dépenses relatives au CPF et combattre la fraude, en effet, les mesures de régulation par la qualité de l'offre du cas du catalogue, le nettoyage des formations, créations d'entreprise et les premières mesures de lutte contre la fraude y ont largement contribué, je pense également à la proposition de loi portée par Monsieur le Sénateur, Martin lévrier qui vise à lutter contre le démarchage abusif et les fraudes qui vous sera bien très bientôt soumise enfin, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais avoir un dernier mot sur la formation aux métiers d'avenir car ce budget encourage l'emploi d'aujourd'hui, mais également de demain pour faire face aux nouveaux enjeux de formation des salariés, le ministère a obtenu une nouvelle enveloppe au titre du FNE, formation et du dispositif Transco à hauteur de 350 millions en autorisations d'engagement et 160 millions d'euros en crédits de paiement en 2023 le FN formation doit permettre de poursuivre l'effort engagé en 2020, 2021 et 2022 afin notamment d'accompagner l'adaptation des compétences des salariés de nos entreprises vers la transition écologique de poursuivent la digitalisation et de favoriser la souveraineté économique et énergétique le dispositif transition collectif permet au salarié qui subirait des courses, les conséquences des mutations économiques de s'orienter vers les secteurs porteurs et aux entreprises dont les emplois sont fragilisés d'accompagner leurs salariés dans dans cette transition en évitant des départs contraints, il y a un enjeu fort à le faire reconnaître par les acteurs et c'est le rôle que nous avons confié au délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles merci à chacun pour le travail que vous avez effectué sur la préparation de ces discussions et je vous propose, effectivement, que nous puissions démarrer le démarrage des discussions, des amendements, merci à tous. Merci madame la ministre, nous allons en effet procédé à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission, je rappelle que pour cette mission, la conférence des présidents a fixé une durée maximum de 2 heures 45, ce qui veut dire que nous devrons avoir terminé à 12

merci Monsieur le Président, alors j'espère, en prenant un peu de la hauteur, arriver à convaincre tout l'hémicycle de l'intérêt de cet amendement, nous convenons tous que la mission Travail emploi s'inscrit dans le PLF 2023 jusque là pas de difficultés, nous avons tous écouté avec beaucoup d'attention le FMI qui nous demande de réduire les déficits publics, nous avons tous écouté avec attention le rapporteur général du budget qui demande à ce que l'État finalement aligne ses propos avec en tout cas soit cohérent avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que dès lors qu'il demande aux collectivités de faire un effort, il s'assigne les mêmes objectifs, à partir de là, et quand on regarde la mission Travail, emploi, alors on peut tordre les chiffres dans tous les sens, ah je vous écouter les uns et les autres, moi quand je suis sur le terrain, je compare BP ABP

ce que propose cet amendement, il propose simplement de réduire, de contribuer à cet effort en réduisant le pic de 500 millions d'euros, ces 500 millions d'euros correspondent exactement à la sous-exécution des 3 premières années et il le conforte également il précise également que nous pourrions effectivement réduire de 300 millions d'euros, le la somme que nous apportons à France compétences alors même que nous laissons un milliard trois pour France compétences alors même que nous venons de mettre en juillet 2 milliards pour France compétences alors même que nouveau n'omettent de mettre en octobre 2 milliards pour France compétences à partir de là, cet amendement et finalement un effort collectif qui est demandé à tous au déficit public et c'est également ah, j'allais dire un amendement de cohérence parce que quand nous sommes sur le terrain et que nous sommes contraints de voter des voter des Budgets que nous avons beaucoup de mal à voter au niveau des collectivités locales, je pense qu'il serait compliqué, très facilement, de laisser passer ces 6 milliards sans un moment donné, contribuer à cet effort de solidarité.

de la dépense et la commission des affaires sociales sur la réduction des dépenses et des crédits, je la partage parfaitement et la commission des finances, partage cet objectif cet amendement présente, à mon avis, 3 inconvénient majeur et manque sa cible première inconvénient, c'est que la commission des finances, a adopté les crédits sans réserve et donc il est en incohérence avec la position adoptée par la commission des finances, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas émis des réserves sur des inquiétudes que nous partageons sur sur le déficit de France compétences mais ça veut dire que nous pensons qu'il faut voter, c'est voter ces crédits tels qu'ils sont, et 2 autres inconvénient c'est que hein, évidemment, il y a des réductions de l'enveloppe liées à l'apprentissage à réaliser, nous partageons aussi cet objectif, les travaux sont commencés la concertation la ministre vient de le rappeler son commencé cependant ça ne portera pas ses fruits cette année puisque que les crédits dans les contrats de cette année qui sont aussi qui seront signés avant la fin de l'année ne sont pas concernés, donc les 300 millions de diminution des crédits pour France compétences sont une mauvaise, une fausse bonne idée, puisque, au contraire, la commission des finances, considère que le fait d'inscrire dès le début 7 milliards en LFI apparaît beaucoup plus sincère, puisque mes chers collègues, il ne faut pas se leurrer, à la fin de l'année les dépenses, elles seront là et ma crainte pourrait tout à fait honnête avec vous, c'est que ce 1,7 milliard ne suffisent pas et la 3ème, raison pour laquelle cet amendement me paraît manquer sa cible, c'est le fait que l'on réduise de 500 millions d'euros, le pique certes les crédits ne sont pas intégralement consommée, mais c'est la fin d'un cycle, nous sommes tous favorables au pic et cela risquerait de pénaliser les conseils régionaux qui sont attributaires en tous les cas qui sont qui ce pic et qui le mettent qui les développent sur le terrain, c'est la raison pour laquelle, c'est une bonne idée, mais il me semble que ça rate sa cible, donc je vous propose, je vous rappelle l'avis de la commission des finances, qui est un avis défavorable. La ville. Alors je rappelle l'avis de la commission des finances, qui vient d'être adopté en commission, ce matin, vous ne deviez pas être là ce matin, mon cher collègue, mais l'avis de la commission des finances, qui a été validé, c'est c'est un avis défavorable. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement, restons calmes. je partage le fait qu'il y a six heures 5 milliards d'euros d'augmentation des crédits de paiement mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, à périmètre constant, c'est beaucoup plus comparables que six heures 5 milliards d'euros, la marche n'est pas aussi haute et et en cela je reprends totalement l'explication qui a été donné par Monsieur Garrido tout à l'heure pour dire que les crédits ne sont pas en augmentation aussi importante que ça, en tout cas, quand on regarde le réalisé par rapport à la prévision pour 2023 surtout 2 éléments sur le fond de l'amendement, d'abord pour ce qui concerne France compétences, nous faisons le choix d'apporter de la trésorerie pour éviter toute forme de rupture, ça ne nous empêche pas de mettre en oeuvre des politiques de rationalisation nous avons conduit la première vague de diminution des du niveau de prise en charge des coûts de formation, nous avons une proposition de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale qui va permettre d'avoir de nouveaux outils de de régulation nous avons prévu et cela fait l'objet d'autres amendements la possibilité d'un d'un ticket modérateur et nous travaillons sur la rationalisation, c'est un chantier suivie par Carole Grandjean tout particulièrement pour faire en sorte d'amener progressivement France compétences à à revenir vers l'équilibre, et nous considérons que la diminution vous proposez pourraient être dangereuses pour la trésorerie de France compétences et le paiement des frais de formation c'est CFA 2ème point concerne le pic, nous avons fait un effort de rationalisation du pic puisque 2023, et de là aussi une année de transition en tenant compte des niveaux de consommation en tenant compte aussi, et d'un engagement pris par le gouvernement il y a quelques mois concernant la reconduction de la totalité des crédits affectés à la part régionale du pic, ce qu'on appelle parfois les prix que vous les pactes régionaux, surtout, nous avons pris connaissance du du rapport du comité scientifique d'évaluation du pic qui montre que le pic permet une augmentation du taux d'emploi 10 points de 57 à 67 % en population générale par les formations qui le permet, il permet une augmentation du taux d'emploi pour les bénéficiaires, qui sont âgés de plus de 50 ans de 33 52 %, ce qui est considérable, c'est une bonne nouvelle, il a permis la l'entrée en formation de 4 1000000 600000 personnes entre 2018 et 2021, ce qui représente une augmentation par rapport à la période 2010 2015 de 460000 personnes formées de plus chaque année et les 2 tiers des entrants sont considérées comme vulnérables au risque de de chômage de longue durée, là aussi c'est une bonne nouvelle et enfin le pic a aussi permis d'augmenter de 100 de 120 à 200000 le nombre de formation pré- qualifiante de préparation des formations qualifiantes pour accompagner les plus éloignés, donc pour toutes ces raisons, l'avis du gouvernement, et est défavorable à cet amendement de de réduction des crédits de France compétences et du pic. je vais demander un scrutin public et monsieur ma chère à la parole pour expliquer son vote. Merci monsieur le président, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors c'est pas tout à fait vrai que la commission des finances, c'est parce que le rapporteur a donné un avis rapidement en tout début de séance que on a passé ensemble des choses, donc faut quand même pas confondre et il ne faut pas trop tordre toujours le règlement parce que sinon, on peut être Captieux, mais c'est pas forcément ce qui est souhaitable je reviens sur les propositions de Frédérique Puissat dans son amendement, que je soutiens évidemment, comme nous l'avons dit dans les interventions du groupe, les républicains, d'une part, il y a des crédits d'en consommer. Donc, ça, il faut quand même en te dire compte un jour dans le vrai budget et après moi j'ai bien entendu pu qui nous dit : mais finalement, il faudra encore en rajouter dans pour France compétences hein, il y a un moment, ça suffit, enfin on ne peut pas continuer comme cela, notamment parce que la vérité, il faudrait peut être la dire aussi sur l'apprentissage, très fortement, c'est que ça profite aux étudiants du supérieur. Et on est en recherche là-dessus de de compétences très vite mais c'est dans le supérieur, que ça profite d'abord oser dire le contraire, il faudra vous le vraiment le prouver avec des chiffres très clair et sur de nombreuses années et on est toujours sur des problèmes qui n'ont pas à avoir avec de l'argent pour les ceux qui sont les moins diplômés, car là c'est bien souvent les normes du travail qui empêche un apprenti de commencer quand vous êtes pâtissier, vous ne pouvez pas commencé quand vous êtes apprenti à 16 ans, à 5 heures du matin, alors alors que les pâtisseries commence à 5 heures du matin, voilà des exemples sérieux et qu'il faut mettre aussi en oeuvre ce n'est pas que du budgétaire, j'en ai bien conscience, je suis sûr que vous allez-y travailler mais en tout cas on ne peut pas continuer à rajouter des milliards et des milliards à France compétences uniquement pour faire plaisir. Je suis donc Monsieur Bruillet, monsieur le rapporteur. je tiens à préciser 2 choses : le la première chose, c'est que c'est un avis des 2 rapporteurs validé ce matin en commission cher Jérôme ma ma 2ème ma 2ème remarque c'est que il y a bien sûr l'apprentissage un bénéfice plus grand pour les catégories de d'étudiants à au niveau de formation, mais il y a aussi un progrès sur l'ensemble des catégories, y compris les bac moins et une reconnaissance de l'apprentissage qu'à mon avis, il convient de souligner et de soutenir ma troisième remarque, c'est pour dire qu'au fond, à titre personnel, je préfère parfois un excédent possible et la sincérité à un déficit masqué. Donc je suis saisi d'une demande non pardon Monsieur Savary. J'ai simplement une réflexion par rapport à l'amendement proposé et ce qui nous a motivés au niveau de la commission des affaires sociales proposer une réduction parce que on est dans un souci d'équilibre budgétaire, hein, et d'ailleurs, le gouvernement semble les semblait partager ce souci puisque Gabriel Attal n'a pas cessé de nous dire de tous les débats de la semaine dernière, ah bah vous faites parfois des dépenses supplémentaires, vous ne me proposer jamais des réductions de dépenses et quand on propose une réduction des dépenses, on nous dit : c'est pas la bonne, alors il faudrait mettre un peu de cohérence dans tout cela et je pense qu'effectivement, si il y a du comparatif compte administratif, comme l'a souligné le rapporteur de la commission des affaires sociales comparatif entre 2022 2023 qui a des possibilités de ne pas tout de suite budgété tout cet effort budgétaire, il sera peut-être éventuellement temps d'y revenir, à travers un PDF rectificatif c'est tout à fait légitime qu'on propose une souche de réduction des dépenses publiques, je tenais à souligner. Donc, cette fois-ci, nous allons procéder au scrutin public, je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, celui du gouvernement, également, il va être procédé au scrutin dans les conditions du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Si le résultat votants 343 331 pour l'amendement 200 Un contre 130 amendement et donc adopté,

ayant vocation à favoriser l'insertion dans l'emploi des jeunes et le retour des demandeurs d'emploi sur le marché du travail y aurait haussant le niveau de qualification, doté de 13 et de 8 milliards d'euros sur la période 2018, 2023 le pic doit ainsi permettre la formation et l'accompagnement de 2 millions de jeunes et de demandeurs d'emploi supplémentaires tout en accélérant par l'investissement, la transformation du système de formation continue, afin d'évaluer la réalisation du pic, un comité scientifique indépendant a vu le jour, doté d'un budget d'un budget de 18 millions d'euros sur la même période, soit 3,5 millions d'euros annuels. Les crédits affectés à l'évaluation du plan d'investissement dans les compétences semblent aujourd'hui disproportionnées, par exemple, en comparaison avec les crédits qui ont été affectés à l'évaluation du plan de relance en effet le comité de l'évaluation du pic et dont est doté d'un budget de 9 fois plus important que celui du plan de relance, ce qui est manifestement selon nous excessif, c'est pourquoi nous proposons un amendement pour un réajustement enfin que les moyens soient affectés au plan d'investissement dans les compétences plutôt qu'à son évaluation merci commission, monsieur le rapporteur. donc il y a un comité scientifique d'évaluation du pic et ce comité vient de rentre d'ailleurs son rapport le 24 novembre dernier je vois vous que je n'ai pas eu le temps d'en prendre totalement connaissance puisque c'était jeudi dernier, la question qui est posée, c'est le coût de cette évaluation de 3,5 millions d'euros, je ne sais pas, pour être tout à fait honnête comment se comment est calculé ce coup

que nous nous exprimons Primon au banc c'est un avis de demande du gouvernement, enfin un avis du gouvernement. Alors Monsieur le Ministre. Mais merci monsieur le président, il s'agit effectivement de 3,5 millions d'euros de crédits pour évaluer 15 milliards d'euros, 3 milliards par an à peu près, en moyenne, donc ça nous paraît être raisonnable en en proportion surtout le travail du conseil scientifique est un travail assez méticuleux, puisqu'il doit examiner non seulement la mise en oeuvre des actions nationales du pic, mais aussi des actions régionales et donc il y a autant d'actions de programmes régionaux que de région, par définition, avec des actions qui sont extrêmement nombreuses et qui nécessite d'aller regarder cordes par Cork les bénéficiaires, l'impact sur le taux d'emploi et et de mener travail rétrospectif et statistiques, c'est la raison pour laquelle, et malgré des efforts qui sont faits par les services en charge le budget de de plus de 3 millions d'euros, 3 millions cinq et et tout à fait nécessaire et ça permet d'éclairer les travaux du Parlement comme du gouvernement avec le rapport du comité scientifique remis chaque année, le rapporteur l'a dit, il a été remis l'année dernière donc demande de retrait sont véritablement des crédits dont nous avons besoin et qui sont utiles pour mener ce vrai travail d'évaluation, y compris pour préparer le le pic post-2023, puisque nous sommes dans une année de transition la transition que j'évoque en 2023 doit nous permet de décider quels sont les volumes que l'on veut investir dans les compétences à partir de 1024. Monsieur Hériot, si il y a une demande de retrait. non, je ne sais pas, demande de retrait, je souhaiterais qu'on puisse voter sur ceux de délibération qui porte sur enfin sur cet amendement, qui porte sur donc une proposition de réduction ou de rééquilibrage, eu égard, encore une fois à l'écart de, de, de l'évaluation qui est porté dans le cas du plan de relance par rapport à cette au pic, donc nous pensons que, il y a vraiment là, on mette en la matière un rééquilibrage à trouver. Monsieur le rapporteur défavorable je mets aux voix l'amendement 66 avec avis défavorable du gouvernement et de la commission qui est pour. Qui est contre. ensuite de 612 présenté par Madame Jasmin, Jasmin qui a la parole. Merci monsieur le président, Monsieur et Madame la Ministre, cet amendement du groupe socialiste vise à rendre effective la 46 jeunes universel. Parce qu'il faut vraiment que ce soit universel en donnant des moyens aux missions locales, d'atteindre l'objectif tous ceux tous les jeunes qui ne sont ni en études ni en emploi ni en formation, soit 1 virgule 5 millions de jeunes, Madame la Ministre, vous venez de dire que vous avez des objectifs ambitieux, donc je crois que cet amendement permettra de prendre en compte l'ensemble des jeunes concernés. En effet, en 2019 un véhicule ces millions de jeunes âgés de 16 à 25 ans n'ont ni emploi ni formation et ne sont pas en sud d'après les données de l'Insee, environ 2 millions de jeunes sans emploi ni formation ni étude n'ont donc pas accès aux si jeune que vous prévoyez, soit 4 jeunes éligible sur 5, dans ces conditions, les effets d'annonce et les effets de langage doit se traduire par la réalité, merci. La commission, monsieur le rapporteur. Qui est pas très clair dans son dispositif, ce que on multiplie par 5 les les moyens alloués aux missions locales, or en réalité de ce que je comprends c'est que ce sont les allocations qu'on voudrait multiplier par 5 le nombre d'allocataires, donc c'est pas tout à fait la même chose que les missions locales, elles, elles accompagnent les jeunes, elle met en place aussi un engagement d'une quinzaine d'heures de travail enfin ou d'activité minimale et puis il y a aussi le le le le bénéfice de la, de l'allocation, mais la l'amendement confond les deux et puis vous l'avez compris de en fait l'idée c'est d'avoir un RSA jeune, or l'avis de la commission est défavorable, sur ces 2,5 milliards.

Abstention : il est pas adopté 610 madame, monsieur Cozic. Merci monsieur le président, donc, cet amendement vise à garantir que les crédits fléchés vers l'indemnisation des demandeurs d'emploi augmente au rythme de l'inflation, en effet, le gouvernement propose une baisse de 21 % des crédits tiennent même action, soit presque 500 millions d'euros supprimer une telle coupe drastique n'est nulle part expliqué dans le projet annuel de performance mis à disposition du Parlement, il convient donc de garantir la stabilité de ses crédits une fois retiré l'effet de l'inflation, telle est l'objet du présent amendement. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Monsieur le Ministre. Des défavorable et la baisse des crédits sur ce programme s'explique par la diminution du nombre d'allocataires de l'ASS, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je ne pense pas que le maintien d'un haut niveau de bénéficiaires de l'ASS soit aussi d'une bonne politique de l'emploi, ce sont des bénéficiaires de l'assurance chômage, en tout cas de l'allocation spécifique de solidarité qu'retourne à l'emploi, donc c'est une très bonne nouvelle et c'est pour ça que nous avons réajusté les crédits en ce sens. Je me vois. Il est retiré, je précise que si ça n'allait pas clair que le précédent n'a pas été adopté ensuite 719 madame, a poursuivi Madame Cohen. Merci monsieur le Président notre amendement d'appel vise à abonder de 200 millions d'euros les crédits pour l'enseignement professionnel public, le président de la République a annoncé la réforme de l'enseignement professionnel, ce qui suscite aussi des inquiétudes légitimes de la part des enseignants qui craignent de voir l'alternance et l'apprentissage de venir la priorité au détriment de l'enseignement professionnel, nous nous refusons cette mise en concurrence, nous pensons que les deux sont nécessaires, mais bien sûr, nous refusons surtout la casse de l'enseignement professionnel qui, comme vous le savez, mes chers collègues, forme les citoyennes et les citoyens donnent des bases techniques solides pour lui substituer, de la formation professionnelle au gré des besoins des besoins des employeurs sans socle théorique, ça n'est pas donc ce que nous défendons et c'est pourquoi nous nous proposons de diminuer de 100 millions euros les crédits pour abonder dans dans le sens de ce que nous défendons, il est bien entendu aussi, et j'en profite, en en défendant ses cet amendement que en général au niveau de mon groupe, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, nous ne sommes pas tellement sur ce jeu d'enveloppe où finalement on retire d'un côté pour alimenter de l'autre, comme si les les les enveloppes sont sont fixées une bonne fois pour toute, c'est un peu un jeu de déshabiller Paul pour habiller Jacques, et c'est vraiment pas dans la conception donc jusqu'à présent, nous ne faisions pas tellement d'amendements en ce sens mais je pense que c'est aussi une façon c'est pour ça que c'est un amendement d'appel d'attirer votre à votre attention sur l'importance de maintenir l'enseignement professionnel, sa qualité et son encadrement. La commission, monsieur le rapporteur. vous l'avez compris c'est un amendement d'appel mais qui ne qui n'a pas lieu d'être, dans nos débats puisqu'il relève pas de la mission Travail, emploi, donc c'est une demande de retrait ou un avis des favoris. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice Cohen, même si je salue l'engagement qui est le vôtre pour accompagner les lycées professionnels et leur réussite et, bien sûr, nous partageons cette volonté, vous le savez, nous sommes en train de préparer aussi les conditions d'une réforme qui donnera tous les moyens au lycée professionnel d'être, d'accompagner la meilleure réussite de l'ensemble des élèves et de favoriser les conditions d'enseignement pour les professeurs, même si nous poursuivons comme vous, cet objectif, il s'agit pour nous de travailler en complémentarité avec la voie de l'apprentissage et la proposition que vous faites au travers d'une mobilité des fonds entre la voie de l'apprentissage et celle du lycée professionnel veux dire, n'est pas pertinent dans la mesure où la voie de l'apprentissage reste une voie de réussite que nous souhaitons continuer à soutenir et nous souhaitons également demain préparer les conditions de la réussite du lycée professionnel vous savez d'ailleurs que dans le lycée professionnel il nous avons 60000 apprentis une augmentation de 42 en 2 ans et que donc l'un et l'autre modèle ne s'oppose pas à notre avis, bien sûr, nous travaillerons demain ensemble sur cette réforme du lycée professionnel, nous avons engagé des discussions avec les partenaires sociaux, des groupes de travail continuons évidemment à construire cette cette cette perspective de réforme qui sera appliqué progressivement et dont l'ensemble des modalités de modalités restent à construire ensemble, aucun avis défavorable, retrait ou avis défavorable. Oui, je veux particulièrement remercier la ministre pour son l'effort d'explication et le fait que ça permet de de montrer quelle est le l'objectif du gouvernement et c'est donc pas une fin de de non recevoir comme nous l'a infligé le rapporteur sans argumentation valable donc non nous allons retirer nos nos notre amendement en attirant quand même toujours votre attention madame la Ministre sur la la la la, l'enseignement professionnel, on le retire parce qu'on sait qu'il sera pas voter, mais voilà les, les choses ont été dites dans l'hémicycle et ça, ça fait valoir notre point de vue. Ensuite, nous avons des amendements en discussion commune, commençons par 611, défendu par Me Jasmin. Merci monsieur le président, au programme accès au retour à l'emploi afin de soutenir l'insertion de l'emploi et l'emploi réellement je dirais parce que le gouvernement propose de diminuer le dans le PLF 2 buts pour 2023 le nombre de Pec, passant de 80000 35000 en 2 ans en 2022, donc c'est une réduction et je crois qu'il faudrait quand même de l'ambition réelle pour en faveur des jeunes. Merci Monsieur le Président, alors effectivement, cet amendement est relatif à cette diminution des parcours emploi compétence, il faut rappeler quand même que lorsqu'on a porté un coup aux contrats aidés en 2018 on a provoqué un vaste plan social silencieux avec la suppression de 250000 contrats et ce, alors même que l'adresse en 2017 écrivait que les contrats aidés permettent de soutenir effectif effectivement l'emploi, voilà que le gouvernement porte un nouveau coup de rabot assez contrats parcours emploi compétence sans que cela nous semble justifier d'aucune manière, il faut mettre fin vraiment au changement intempestif concernant la prise en charge, notamment dans certaines régions en Île France par exemple, en mars dernier l'arrêté préfectoral limitait les possibilités de renouvellement à 6 mois et le taux de prise en charge à 40 pour 100 45 %, un coup de canif énorme pour les acteurs dans l'Ardèche, la transformation des contrats aidés en parcours emploi compétences et s'est accompagnée d'une baisse de 72 % du nombre de contrats entre 2017 et 2018 en 2022, nous sommes donc à 67000 bénéficiaires en parcours emploi compétence au total, ce qui est peu compte tenu du nombre de personnes éloignées de l'emploi dans le pays et du nombre d'acteurs collectivités ou associations qui peuvent accueillir et qui peuvent, par aussi bénéficier d'un appui via ce ce dispositif, il faut donc faire plus en conséquence, nous proposons d'allouer les 150 millions d'euros, qui correspond tout simplement au maintien pour 2023 des paramètres appliquée en 2022 concernant ces ces contrats et donc, à savoir 100000 emplois pour une durée totale de 24 mois renouvellement inclus et taux de prise en charge compris. L'avis de la commission monsieur rapporteur. Merci monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur la réponse qui m'a été faite tout à l'heure par Madame Cohen, ça n'est pas du tout. Un manque de respect vis à vis de la question qui était posée, le fait que j'ai renvoyé au ministre mais en fait il se trouve que je suis rapporteur spécial du budget, travail, emploi et les crédits dont vous solliciter l'augmentation sont des crédits de la mission enseignement supérieur auquel je ne connais rien donc je préférerais que ce soit, Madame la Ministre, qui répondent et qui vous apporte la réponse complète, et ce d'autant plus que nous sommes dans un temps contraint donc n'y voyait pas une forme de, de, de désinvolture de ma part ou de désintérêt, c'est juste que je souhaitais que vous ayez une réponse complète et charpentée que je ne suis n'était pas en mesure de vous apporter pour ces 2 amendements, c'est un avis défavorable pour la raison suivante les buts, de cette année, prévoit un maintien des entrées en contrats aidés dans le secteur non marchand, donc les femmes au même niveau que 2022, avec une diminution portant sur les contrats dans le secteur non marchand, qui ne sont pas visés par votre amendement la relance des contrats aidés est intervenue dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, la situation aujourd'hui objectivement n'est plus la même et traditionnellement, la commission des finances est assez réservé sur ce type de dispositif donc l'avis est défavorable sur ces deux amendements qui visent à augmenter de 150 millions d'euros, la dotation pour les contrats aidés.

On ne parlera plus beaucoup après monsieur le président, puisque de toute façon c'est con, c'est c'est comme vous l'avez dit, contraint par des horaires voilà sur les contrats aidés sur les contrats, excusez-moi, sur la proposition qui est faite par nos collègues, nous allons soutenir, même si dans mon groupe, nous pensons que les contrats ne sont pas la panacée, parce que ce qui peut régler le problème aujourd'hui est bien des gens les plus éloignés de l'emploi, ce sont de véritables formations et de véritables emplois et non pas des petits contrats qui finalement s'arrête un jour ou l'autre, ceci dit, ça a été dit, on a supprimé les contrats aidés aujourd'hui les Budgets alloués par l'État à Pôle emploi ont été dit suspendu, notamment les contrats APEC pour les municipalités, nous avons été interpellés par de nombreux maires qui, du jour au lendemain, ont été avertis que leur contrat été interrompu et pour les petites communes, il faut bien se le dire, c'est un coût supplémentaire, Je pense que ces contrats avaient un intérêt lorsque ces gens se retrouver dans les municipalités, c'est qu'ils pouvaient bénéficier d'une formation et d'un retour et d'un et d'un retour peu à peu à l'emploi puisqu'on leur permettait de se remettre le pied à l'étrier et donc pour ces raisons, même si nous pensons que la formation est essentielle, nous allons soutenir les amendements de nos collègues. Je mets aux voix donc, pour commencer, l'amendement 611 avec double avis défavorable qui est pour. Contre. Abstention est pas adopté sur le 660 même vote même vote pas adopté, non plus, amendement 606 monsieur le mien. Merci monsieur le président, donc, cet amendement est relatif oppose insertion dans les ateliers chantiers insertion en effet ces ateliers salarie et accompagne chaque année environ 165000 personnes ce qui représente plus de la moitié des effectifs de l'insertion par l'activité économique, or le budget 2023 prévoit une diminution de 6 % du nombre de postes dans ses ACI c'est regrettable parce que, d'une part les ACI ont démontré leur capacité de développement avec une croissance de près de 30 % des contrats signés entre 2018 et 2022, et d'autre part, comme chacun le sait, il s'adresse aux personnes les plus éloignées de l'emploi, c'est pour ça que par le pardon, par le biais de cet amendement, nous proposons de mobiliser pleinement la capacité des ateliers et chantiers insertion a accompagner vers et dans l'emploi les personnes qui en sont le plus exclus, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, alors c'est le 1er Ramon demande une série assez importante d'amendement qui vise à majorer les crédits destinés aux structures d'section l'insertion par l'activité économique est incontestablement une forme extrêmement pertinente d'accompagnement vers l'emploi, notamment pour les demandeurs d'emploi de très longue durée des bénéficiaires du RSA ou des jeunes très éloignés de l'emploi. Les crédits sont en légère progression en 2023 et les structures aurait sans doute souhaité disposer d'une marge budgétaire plus importante, d'où cette série d'amendements toutefois le secteur, je vous le rappelle, a été extrêmement soutenue ces 4 dernières années, les crédits était 840 millions en 2018 et de 900 millions en 2019, ils sont passés à 1 virgule 3 milliards en 2023, c'est une augmentation de l'ordre de 50 % sur les 4 dernières années, compte tenu de cette progression sur 3 ans du niveau de consommation de crédits en 2022, qui est d'environ 1,2 milliards de la légère augmentation cette année, et par ailleurs de l'effort budgétaire dont nous parlons beaucoup depuis le début de cette matinée, il me semble qu'il n'est pas. Souhaitable d'aller au-delà de la dotation prévue pour 2023 donc c'est donc un avis de retrait ou un avis défavorable. Merci monsieur le président, c'est c'est un avis défavorable, comme cela a été dit, les crédits liés à eux, ont augmenté de 400 millions d'euros depuis 2018, ils atteignent à nouveau un montant record à plus d'un milliard 300 millions d'euros, c'est la première fois que nous atteignons autant de de soutien à l'IAE, l'objectif reste le même : atteindre en 2025, 122000 ETP, soit à peu près 140000 personnes qui ou qui pourront être accompagnés en matière d'IAE et avec une trajectoire de montée en puissance qui tienne compte aussi de la réalité et la réalité c'est que ses propres ses structures d'insertion rencontre aussi des difficultés de recrutement, et donc le budget que nous prévoyons, est en hausse, il permet d'absorber l'augmentation du SMIC et permettra de créer 5 à 7000 postes de de financer 5 à 7000 postes de plus 2022, non pas par rapport à la prévision 2022, mais par rapport à ce qui sera réalisé puisque à date, nous savons que les crédits prévus pour 2022 en matière de financement des postes ne seront pas tous consommés et que l'objectif en terme de poste ne sera pas atteint donc par rapport à ce qui est réalisé en 2022, nous serons en augmentation de 5 à 7000 postes donc défavorable.

Merci monsieur mini et le président, cet amendement vise à créer un programme spécifique pour la santé mentale et particulièrement la santé mentale des travailleurs, la France se caractérise par un déficit de reconnaissance des maladies psychiques au travail comme maladie professionnelle, alors que la loi numéro 2015 en tirer 9194 du 17 août 2015 relatives au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen dispose bien les les maladies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, le coût économique de ces maladies entre un véhicule 9 à 3 milliards d'euros par an est élevé et nous constatons qu'il y a pas beaucoup d'effet par ce gouvernement pour cette prise en compte, donc nous voulons créer ce programme avec des fonds disait et dédié à la santé mentale des travailleurs, un fonds de 100 millions d'euros avec une autorisation d'engagement des crédits de paiement, je souhaite vraiment cher collègue que vous puissiez prendre en compte cette situation merci. vous l'avez compris qui vise à créer un nouveau programme avec un fonds dédié à la santé mentale, doté de 100 millions d'euros. Donc, cet amendement est est assez compliqué parce que c'est compliqué de faire le rapport entre le constat qui est fait entre cette difficulté que nous avons à reconnaître davantage les maladies mentales dans l'entreprise avec le fait que l'amendement lui- même constate qu'il y a de plus en plus de reconnaissance en maladies professionnelles des maladies de des syndromes notamment onction dépressif, cependant je vous vois pas bien en quoi la création d'un fonds de 100 millions d'euros pourrait améliorer notamment ce qu'indique le le le le l'amendement les sanctions à l'égard de ce type de comportement donc j'entends le sujet, j'entends la politique qui peut être menée pour renforcer la lutte contre les maladies professionnelles et notamment les maladies mentales, mais quel type d'action financerait ces 100 millions demandés il me semble que l'exposé des motifs reste extrêmement flou sur la question et c'est donc un avis défavorable. Merci monsieur le président, madame la sénatrice, nous partageons l'enjeu autour de, de, de la prise en charge de la santé mentale et d'une meilleure prévention et pour cela le le gouvernement est pleinement engagé pleinement engagé déjà par l'engagement pris et le travail effectué par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui ont publié des guides pour effectivement accompagner cet enjeu mais je voudrais rappeler également, et, et, vous le savez, pour cause, le le la loi du 2 août 2021 qui vient améliorer la prévention en santé au travail et qui a largement accompagné ce sujet là, notamment entre autour du rendez-vous de liaison des services de prévention santé au travail de la lutte contre la désinsertion professionnelle et d'un certain nombre d'outils qui viennent, accompagné notamment cet enjeu de la santé mentale et ça a fait l'objet lors des discussions parlementaires d'un attachement fort de l'ensemble des parlementaires des 2 chambres pour que cet enjeu-là soient bien pris en compte dans les dans le renforcement de la prévention en santé au travail et puis je voudrais rappeler aussi le travail des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui a été renforcée est terminée aussi par le vous rappeler le le le 4ème plan santé au travail, qui depuis décembre 2021 ah là aussi renforcer un certain nombre d'axes, notamment celui des TPE-PME qui ont été mieux outillée pour qu'il développe des outils pour travailler sur les risques psychosociaux qui a également prévu de faire une meilleure prévention pour le secteur agricole, dont on sait que les enjeux en santé au travail sont extrêmement importants, a également prévu de mieux des consultants pour accompagner cet enjeu là et a souhaité développer aussi l'accompagnement lors de d'évolutions organisationnelles des entreprises pour accompagner l'enjeu de la santé au travail avec une dotation exceptionnelle de 2 1 millions d'euros, je tiens à le rappeler, donc je crois que cet enjeu-là et est d'ores et déjà 13 accompagné très suivie et c'est un axe évidemment que nous partageons avec vous année, je mets aux voix l'amendement 614 avec 2 avis défavorable qui est pour. Je parle des pour l'amendement 614 avec double avis défavorable qui est pour.

Merci monsieur le Président notre un moment et donc un amendement d'appel qui vise à renforcer les crédits de l'inclusion par l'activité économique de 100 millions d'euros afin d'augmenter le nombre de postes consacrés à ce secteur en 2023 si le gouvernement veut atteindre le plein emploi, il faut mettre les moyens à la hauteur de ses ambitions en s'adressant à celles et ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail, le secteur de l'insertion par l'activité des entreprises représentaient est un secteur en dynamique portée par les entreprises d'insertion, des entreprises de travail temporaire d'insertion et les entreprises d'insertion par le travail indépendant notre amendement vise donc à envoyer un signal de soutien à ce secteur, je vous remercie. Madame la rapporteure de la commission affaires sociales. Oui, merci Monsieur le Président, je vais défendre l'amendement de mon collègue Philippe mouiller qui n'a pas pu être présent, alors il pèse un peu moins que celui de. Question une attendu une seconde.

que celui de notre collègue puisqu'il pèse effectivement 30 millions d'euros, c'est, c'est vrai, Monsieur le Ministre, que je, je crois qu'on est tous attachés à la aux structures d'insertion par l'activité économique et que les gouvernements précédents ont fait un effort considérable sur les à eux, on a eu un texte de loi, il y a pas très longtemps dans cet hémicycle, je crois que personne ne doute de nos intérêts sur sur ces outils-là, par contre, quand on regarde quand même les chiffres avec précision, Monsieur le Ministre, on s'aperçoit quand même que même en considérant la sous-consommation 2022 que vous avez évoqué un mettre 1,27 % de plus au global ne rattrape pas la hausse unitaire de 9,5 % à partir de là, les structures ont 2 solutions : soit, effectivement, elles arrêtent de faire des contrats, soit elle privilégie elles-mêmes un certain nombre de contrats plutôt sur ce qui est peu coûteux d'ailleurs les associations intermédiaires et non pas les chantiers d'insertion, moi je considère, nous, nous considérons que ce ne sont pas aux structures de faire ses choix mais c'est un choix politique, donc 2 possibilités : soit on fait un choix politique qui ont dit on met plutôt l'accent sur les associations intermédiaires, du coup, on suit pas forcément les besoins du terrain : soit on fait une rallonge de or de 30 millions d'euros, c'est ce que nous vous proposons dans cet amendement. Nous avons un 2ème amendement identique 488 monsieur Boyer ses collègues Alain pensait manger. Merci monsieur le président, alors le gouvernement effectivement nous nous annonce le retour au plein emploi, il nous semble indispensable que cette amélioration profite aussi à ça des ceux des plus éloignés du marché du travail, pour cela, donc nous proposons comme il a été dit soutenir l'insertion par l'activité économique en prévoyant budgétairement davantage en 2 2023 en effet, si le budget présenté pour 2023 est en augmentation en valeur, il est en réalité en diminution au nom d'été d'équivalents temps plein finançable, compte tenu de la hausse du SMIC, vous savez que la loi prévoit en effet que les montants unitaires des aides au poste sont indexés sur le SMIC aussi cet amendement permet de poursuivre la dynamique du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique et aussi je vous propose de préserver cette dynamique de l'effort budgétaire, car c'est un investissement. Même même avait amendements identiques Monsieur Jomier. Oui merci monsieur le président, j'ajouterai juste quelques mots, c'est que si le budget effectivement en augmentation

par ailleurs, la loi prévoit que les montants unitaires des aides au postes sont indexés sur le SMIC, d'où la nécessité de majorer de 30 millions cette ligne. Maintenant la ville, la commission d'une part sur le 717 et ensuite sur les trois amendements identiques. Alors l'avis de la commission, je l'ai déjà donné tout à l'heure sur l'ensemble des des amendements de ce type, c'est un avis défavorable sur les quatres avec évidemment un regard plus spécifique sur les trois amendements identiques mouillé Breuiller et Ferret, qui sont évidemment extrêmement sympathique et généreux mais faut quand même qu'on n'oublie pas et c'est le rôle de la commission des finances, on a dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention aux dépenses publiques, qu'il fallait réduire même le budget de la mission Travail et emploi, on ne peut pas, de l'autre côté, répondent à une demande qui est tout à fait légitime de de des acteurs de l'insertion par l'activité économique qui font un travail travail formidable, mais qui ont vu leur budget progresser de façon très très sensible à ces 4 dernières années, ça été rappelé par le ministre tout à l'heure, plus 400 millions d'euros sur les 4 dernières années, le budget augmente cette année également, à peu près 16 millions d'euros de de mémoire, ça ne couvre sans doute pas, effectivement, l'inflation, mais au titre de la commission des finances, je ne peux pas donner un avis favorable.

a pu, a bien donner l'avis de la commission, il tient aussi à on a parlé de santé mentale à à éviter le risque de schizophrénie pour les rapporteurs, le rapporteur spécial que je suis et qui a signé un des amendements juste pour souligner que cet amendement était très débattu et il a donné le résultat de la commission. ce policier. Nous allons retirer notre amendement pour donner plus de poids à ceux de nos collègues qui demande un peu moins mais bon voilà, on va être raisonnable.

Merci monsieur le Président, pour un montant de 81 1000000 817070 euros, il s'agit de maintenir une qualité de l'accompagnement mis en oeuvre dans ces différentes structures merci.

Oui, hé bien, cet amendement du groupe socialiste vise à développer la formation dans les il y a le budget de formation pour l'insertion par l'activité économique est porté à 100 millions d'euros en 2023 oh c'est du plan d'investissement dans les compétences en augmentation de plus de 25 % par rapport à fin 2022 donc il s'agit maintenant de prendre en compte les nouveaux besoins pour permettre la réalisation de toutes les formations dans ce cadre, je vous remercie.

l'expérimentation territoire zéro chômeur conduite entre 2016 et 2021, est un dispositif dynamique qui a permis à plus d'un millier de personnes éloignées de l'emploi, de retrouver du travail, 50 nouveaux territoires peuvent désormais lettre entre juillet 21 et juillet 2024 sachant que l'association pense être en mesure de couvrir 60, territoire d'ici 2023 ah si afin que cette expérimentation qui, rappelons-le, permet le retour à des emplois en CDI des emplois à la forte utilité sociale et environnementale donc répondant à l'aspiration d'y trouver du sens et qui participent au dynamisme des territoires puissent vraiment se déployer il faut que les crédits alloués soit suffisant dès lors par cet amendement, nous souhaitons augmenter les moyens dévolus aux expérimentations territoires zéro, chômeur de longue durée, en vue notamment de l'augmentation du nombre de territoires habilité afin qu'aucun projet mature ne se voit refuser par manque de crédit. merci. Et l'avis de la commission. ces crédits ont déjà progressé notablement en 2023 puisqu'il passe de 33 à 45 millions d'euros avec l'amendement serait ce serait donc une multiplication par 3 sur un an, je ne suis pas certain, même avec l'extension à de nouveaux territoires volontaires qu'une telle montée en charge soit réaliste, compte tenu du niveau constaté des embauches dans les entreprises à but d'emploi depuis le début de l'expérimentation dont tout le monde se satisfait sur le terrain mais le le le l'enjeu paraît un petit peu fort pour cette année.

merci Monsieur le Président, dispositif de cohérence également parce qu'il y a beaucoup de chômage et quand on prend des mesures pour essayer de trouver des solutions, y compris pour les structures d'accompagnement de nos jeunes, hé bien, on voit que rien n'est adoptée et là ça me suis point considérablement merci. Retrait ou défavorable, je précise qu'on a déjà augmenté de 30 millions d'euros tout à l'heure, donc là c'est c'est 20 millions mais complémentaires. Monsieur le même avis,

merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, comme j'ai déjà développé l'argumentation en faveur de cet amendement dans mon dans mon intervention de tout à l'heure je ne développe pas, mais il s'agit de proposer une augmentation de 5 millions d'euros pour

même, c'est le même un amendement que celui de de nos collègues centristes, donc effectivement, nous trouvons que c'est tout à fait dommageable de mettre en danger un outil qui est précieux sur les sur les territoires, et d'ailleurs, un outil pour lequel les maires sont particulièrement attachés, c'est important d'avoir un un lien de proximité avec les personnes qui sont éloignées de l'emploi et et donc c'est pourquoi nous nous faisons cet amendement, je vous remercie. l'avis de la commission. par amendement, cette hausse de 5 millions que vous sollicitez donc en réalité, cet amendement est satisfait : c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne l'ai pas déposé cette année, comme je le déposais d'habitude chaque année comme vous, mes chers collègues, donc il est satisfait, c'est donc une demande de retrait. c'est le même avis, pour une raison qui m'échappe un peu, monsieur le président, le financement des maisons de l'emploi et systématiquement pourvu par amendement parlementaire et et rarement dans la maquette initiale du PLF nous avons reconduit cette tradition, mais comme l'a dit le le rapporteur à l'instant, l'amendement du rapporteur spécial de l'assemblée nationale telle qu'il a été intégré à l'occasion de l'engagement du 49 3 permet de satisfaire les 2 amendements qui sont déposés, donc si demande de retrait. Demande de retraite retiré.

Abstention est pas adopté. Nous avons quatre amendements discussion commune, commençons par le 616 madame Vogel. Si monsieur le président, cet amendement propose d'évaluer les coûts et les modalités d'adaptation du monde du travail à la crise climatique, nous ne savons toutes et tous, le réchauffement climatique est déjà là, et si nous continuons sur la même trajectoire, il fera en moyenne 3,2 degrés de plus d'ici la fin du siècle, et quand bien même nous prendrions des aujourd'hui les décisions nécessaires pour éviter la catastrophe, certains impacts de la crise climatique sont irréversibles et face à ces derniers, il y a pas le choix, il faut nous adapter dès maintenant et notamment adapté le monde du travail avec une simple hausse des températures mondiales de 1 virgule 5 degrés qui, elle, malheureusement, est inéluctable, plus de 20 millions de travailleurs seraient exposés chaque année un risque de décès en raison d'une chaleur excessive de 2 pour 100 des heures de travail annuel pourrait être perdus mondialement le boum de l'utilisation de la climatisation que nous avons vu cet été et plus qu'une impasse c'est un accélérateur de la crise, c'est donc vers d'autres changements qu'il faut aller sur les horaires de travail sur les rythmes, sur l'année sur les tâches, les lieux de travail leur adaptabilité aux vagues de chaleur pour cette raison, une des propositions du rapport sénatorial dont j'ai eu l'honneur d'être le rapport triste sur la sécurité sociale, écologique était d'évaluer la prévalence des pics de chaleur dans les années à venir, afin d'acc d'encourager les employeurs et employeuses à y préparer afin de préserver la santé des travailleurs et des travailleuses, cet amendement ne fait que refléter cette proposition et propose donc des fonds pour une étude dédiée à l'évaluation des coûts et des modalités d'adaptation du monde du travail de demain à la réalité du réchauffement climatique et évidemment, nous demandons au gouvernement de lever le gage.

vice-vise donc à augmenter de 4 millions d'euros en 2023, les crédits de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, ces dernières années, l'AFPA a subi des diminutions successives du nombre d'emplois ainsi la loi de finances pour 2022 a réduit de 94 équivalents temps plein travaillés le plafond d'emplois de l'AFPA dans ce PLF pour 2023, le poids, le plafond d'emplois est fixé à 5487 E ETP, ce qui représente une nouvelle diminution de 61 par rapport à 2022, et nous le regrettons cette politique d'austérité à l'égard d'un opérateur qui a déjà vu ses effectifs diminuer dans des proportions significatives au cours des dernières années ne paraît évidemment pas justifié le projet annuel de performance de la mission Travail et emploi prévoit que l'année 23 sera, je cite, malgré marquée par plusieurs chantiers d'importance sur la stratégie globale de l'établissement public et la politique de certification professionnelle que l'Agence conduit conduit pour le ministère du Travail, ce qui a été décidé, je cite encore de lui transférer plusieurs missions sur la politique du titre professionnel du ministère du Travail aujourd'hui assurées par les services déconcentrés pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de maintenir le plafond d'emplois à son niveau de 2022 telle et le sens de l'amendement. Et enfin, dans les discussions, quand même Madame projet vous avez 2 autres amendements si 19 et 621. Merci monsieur le président, leur le 619 très ah le le l'étude sur un congé parental égal en France, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des espèces de la société, très loin d'être atteinte et en particulier au niveau des salaires et de la charge parentale, un des événements majeurs qui structure cette inégalité, c'est l'arrivée d'un premier enfant dans un couple hétérosexuel, la charge de la parentalité revient majoritairement à la mer, affectant durablement sa carrière et conditionnant un rôle social au sein de la famille, et plus largement au sein de la société, l'existence de cette inégalité, elle est favorisée encouragée construite par notre société, qui attribue à la mère qui a accouché principalement et de façon totalement disproportionnée par rapport au père ou au deuxième par an, la charge de s'en occuper, après la naissance, via un congé par parentalité absolument inégalitaire, en effet, bien que le congé paternité était un peu allongé, il demeure plus court que le congé maternité sans aucune justification et de nombreux pères ont des difficultés pour l'obtenir auprès de leur employeurs et employeuses conséquence si son salaire était déjà en fait inférieur à celui de son conjoint ou s'il était à peu près similaire, les études démontrent que ce n'est plus le cas, ensuite pour la mer, par ailleurs, l'inégalité entre les deux parents vis-à-vis du congé parentalité crée une forte discrimination à l'embauche, puisque les employeurs savent qu'une femme en âge de procréer pourrait partir en congé maternité et que ce risque est presque nulle en cas d'embauche d'un homme en âge de procréer, il n'y a pourtant aucune raison qui puisse justifier si l'on reconnaît qu'un enfant a 2 parents de ne pas reconnaître le même congé pour les 2 parents, la seule manière d'assurer l'égalité, c'est d'avoir un congé parentalité égal et obligatoire, il existe plusieurs modèles dans le monde, comme en Suède ou en Espagne, et je vous propose simplement d'étudier simplement d'étudier comment nous pourrions instaurer un congé parental obligatoire de cette semaine pour aller vers une société plus égalitaire, je vous remercie. L'autre n'a rien à voir. Donc, le 621 maintenant, c'est un amendement qui vise à étudier la mise en place d'un congé menstruel, alors je ne vous apprends rien quand je vous dis que la moitié de la population française environ a eu ou aura ses règles ou aura ses règles pendant environ 38 ans de sa vie, cette réalité objective de la vie de la moitié de la population, 3 jours par mois pendant à peu près la moitié de sa vie est entouré d'un tabou, on ne dit pas qu'on a ses règles, on se passe des tampons discrètement comme c'était une honte, et on ne traite pas socialement le fait que les règles impacte nos vies peuvent engendrer des douleurs, des effets objectivement handicapant pendant quelques jours pour travailler certaines femmes et personne monstrueux ont le sentiment qu'on leur enfonce des clous dans le ventre, qu'on leur coupe les organes ont des bouffées de chaleur, maux de tête, des vertiges etc alors parfois il s'agit des effets secondaires de l'endométriose oui puis parfois pas personnellement, j'ai parfois tellement mal que je peux pas me lever, mais j'ai pas d'endométriose, or la société ne prévoit pas de gérer cette réalité, le monde du travail a été fabriqué par des hommes pour des hommes et les femmes s'emploie à ne pas faire exister une spécificité de peur d'être discriminé alors beaucoup d'adaptations sont à faire pour prendre en compte le fait que les menstruations existe, l'une d'entre elles qui doit venir dans un ensemble de mesures, c'est le congé menstruel je vous propose d'ne réfléchir à sa création, en Espagne, il est possible de prendre 3 jours de congé cinq en cas de symptômes aigus en France, plusieurs entreprises ont choisi d'expérimenter avec succès ce dispositif, ce qui va dans le bon sens mais il faudrait qu'ils soient étendues afin de couvrir toutes les personnes concernées, d'autant que je vous le rappelle 68 % des Françaises sont en faveur un congé menstruel. Alors, sur ces quatre amendements messieurs rapporteur l'avis de la commission. Oui, monsieur le Président, très rapidement, sur ces quatre amendements qui sont en discussion commune mais qui n'ont en commun que le gage, puisque vous avez compris qu'on touche à quatre sujets extrêmement variés dans l'ordre, donc le changement climatique un avis, c'est une demande de retrait ou sinon un avis défavorable sur le la transition écologique, ça fait partie très clairement des axes de travail de l'Anact, donc de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, donc il ne nous semble pas opportun de créer un fonds spécial d'adaptation qui serait crédité de 5 millions d'euros pour l'AFPA c'est également un avis de retrait ou défavorable puisque l'AFPA est fortement soutenu par l'État et a bénéficié d'une subvention complémentaire en PLFR et elle doit continuer à se restructurer sur les deux derniers amendements où notre collègue ah les a même interverti

on comprend bien l'idée, ce sont des sujets qui dépassent largement les compétences de la mission Travail emploi hein et et qui font plus l'objet de débats sociaux, sociétaux, je dirais, qui sont tout à fait important, il me semble pas que l'étude d'une nouvelle évolution législative parce que c'est une nouvelle et tu es législation qui est appelé de vos voeux rentre dans les demande des crédits supplémentaires, ça rentre dans les, dans les fonctions et dans les crédits inhérent au ministère du Travail à la délégation générale au travail, la direction, pardon, de telle sorte que joue dans son demande le retrait. L'avis du gouvernement, donc je vais mettre aux voix successivement ces quatre amendements avec un avis de retrait ou défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement, commençons par l'amendement 616 et pour. Qui est contre. L'abstention est pas adopté, amendement 716 également avis défavorable et le gouvernement même faute. Amendement 619 même vote et s'en il a toujours même vote. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission donc travailler emploi n'est pas une demande d'explication de vote, je rappelle que la ville de la commission est favorable de la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de la mission, je le mets aux voix mais j'ai une demande de scrutin public du groupe, les républicains sur la mission avec un avis favorable de faire de la de la commission, il va être procédure au scrutin public dans les commissions sur les

Ne demande à voter, le scrutin est clos. Voilà le résultat votants 343 331 pour les crédits 240 contre 91 ans que les crédits sont adoptés sont adoptés encore à discuter les articles rattachés à la mission article 47, je le mets aux voix qui est pour. Contre il est adopté, article 48 jeunes mais également voix qui est pour. Contre, abstention il est adopté à l'article 49 j'ai trois amendements en discussion commune commence par madame Lavarde 678. Oui, merci Monsieur le Président, alors en fait cet amendement suit exactement la même logique que ceux qui ont été déposés par les les 2 rapporteurs, sauf qu'il va plus loin puisque l'amendement des rapporteurs prévoient la possibilité de moduler le prix pour certaines formations et donc moi mon amendement prévoit en fait un plafonnement pour toutes les formations et introduit aussi un ticket modérateur alors pourquoi, parce que, enfin moi je pense que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc si on veut vraiment engager pleinement les gens dans un processus de formation et que ce soit pas la réponse à un coup de fil, on leur dit : vous avez un compte, n'oubliez pas d'utiliser vos crédits ben si on les fait participer un peu, on est certain un gros seront et qui seront vraiment acteurs de cette formation et bien évidemment, l'idée n'est pas de faire payer ce ticket modérateur à tout le monde quand tu la formation elle s'inscrit dans une procédure de retour à l'emploi dans une procédure de réorientation professionnelle, là il n'y a pas lieu d'être, parce qu'on est vraiment dans un accompagnement vers le marché du travail, mais par contre pour toutes les autres formations qui, parfois, peuvent être des formations, pas de confort, mais peut être un peu moins engagé, il me semble qu'il est vraiment utile d'introduire ce plafonnement et ce et ce ticket modérateur. Ensuite, monsieur le rapporteur, kaput et madame la rapporteure, puis ça vous présentez vos amendements. Alors merci Monsieur le Président, donc on a un amendement de la commission des finances, qui a été travailler avec la commission des affaires sociales qui vise le même objectif de régulation mais qui est plus raisonnable et plus limité, de façon moins budgétaire, je vous rappelle que l'augmentation forte et non maîtrisée, les dépenses induites par l'utilisation du CPF, justifie la mise en place de mécanismes de de régulation, c'est ce qui est prévu par l'article 49 du gouvernement nous souhaitons juste au, comment élargir ce mécanisme de régulation en prévoyant qu'un plafonnement soit possible, nous n'allons pas jusqu'à faire ce que sollicite madame Lavarde comme ça, je défends je, je, je donne mon avis en même temps et c'est la c'est la raison pour laquelle je lui demanderai de retirer le sien au profit de l'amendement de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, parce que l'objectif n'est pas de mettre un ticket modérateur ceux qui ressortiraient de l'amendement de Madame Lavarde, de la façon dont il est rédigé. Madame la rapporteure de la commission. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, simplement rappeler la mission que nous avions conduit avec Martin lévrier Corinne Ferré, qui consiste effectivement à ce qu'on ait un reste à charge pour les personnes qui faisaient des formations avec un objectif de recentrer le CPF sur l'employabilité d'utilisateur et sur le développement des compétences infidélité professionnelle en ce sens ont rejoint tout à fait les objectifs de Christine Lavarde qui, je le comprends, hein, à une vision budgétaire de ce qui se passe sur France compétences parce que je pense que les PLFR à 2 milliards qui nous arrive régulièrement commence à vraiment nous poser question sur notre capacité à équilibrer France compétence donc bien entendu que je je défends le l'amendement que nous avons posée mais je comprends tout à fait la position de Christine Lagarde. Qu'est l'avis du gouvernement Madame le rapport de Madame. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, effectivement, même avis que la commission au fond le le l'enjeu effectivement est d'accompagner le le compte personnel de formation maintenant dans un degré de maturité si le CPF est un vrai succès avec 5,5 millions d'ouverture de ses comptes de formation qui ouvre l'accès aux droits à formation et à la mobilisation de ses droits à formation c'est un vrai succès, c'est un vrai succès populaire que nous souhaitons bien sûr accompagné néanmoins nous avons évidemment le partage avec vous de cette profonde conviction et de cette nécessité d'avoir un mécanisme de régulation pour que ces fonds soient mobilisés à des fins d'employabilité et de maintien dans l'emploi d'accompagnement des compétences sur des projets professionnels et donc c'est là je reviens l'objet du du de la proposition d'amendement pour le ticket modérateur,

cette orientation sur un projet professionnel solide donc un avis défavorable à cet amendement. Et sur les deux amendements identiques, je vous, je vous demande aussi l'avis du gouvernement sur les 2 autres. 28 et 376 sagesse. Madame Lavarde je vous avez une demande de retrait, qu'en pensez-vous. Ah non, mais j'ai peut-être une lecture trop budgétaire mais moi je vais laisser mon amendement juste quand même pour Monsieur kaput c'est les modalités des 2 dispositifs sont définies par décret, donc ça ne veut pas dire que ce sera obligatoire pour tout le monde, et j'entends la Ministre dire qu'elle est prête à faire des réformes, mais surtout n'allons pas trop vite, enfin je veux dire à chaque fois qu'on fait un texte budgétaire on rajoute en gros 2 milliards sur France compétences alors je veux bien que les milliards pleuvent, mais il faut vraiment engager ce sujet et là ce que je vous propose, c'est de le faire et ensuite par décret, bien évidemment, de choisir les cas de figure, où le plafond ou le ticket modérateur, n'a pas raison de s'appliquer, mais pour tous les autres, enfin, sinon on va continuer à être harcelés au téléphone et puis le jour où on a de l'argent, dira oui, Givet et puis quand on en a pas assez Bandiera malheureusement je peux pas aller faire cette formation mais peut être demain, dès que j'aurai acquis à ces droits, donc là, voilà, c'est juste un pour essayer vraiment de rentrer dans ce sujet. Monsieur le Ministre. Simplement, monsieur le président, pour pour dire madame la sénatrice Lavarde que la la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale que vous aviez examiner interdira, purement et simplement le démarchage téléphonique, ce qui est une bonne chose et et traitera le sujet par d'autres aspects, je crois qu'avec la rédaction qui soit là qui la vôtre, le décret ne puisse plus permettre justement une exonération totale de ticket modérateur, ce qui serait problématique, par exemple pour les demandeurs d'emploi de très longue durée qui, confronté à des difficultés financières ne pouvaient plus accéder à l'information, et donc il y a vraiment on vraiment une difficulté avec la rédaction, qui est la vôtre, raison pour laquelle le gouvernement préfère d'où la vie de sagesse exprimer par Madame la Ministre, les amendements 28 et 376. Alors je mets aux voilà une maman 678 de madame Lavarde avec vide retrait ou défavorables des de de la commission du gouvernement qui est pour.

Abstention : ils sont adoptés. Je mets donc aux voix avec cet amendement à l'article 49 modifié qui est pour l'article. Attention, il est adopté, mes chers collègues, nous avons tenu finalement l'horaire au regard du nombre d'amendements à examiner sur la Solidarité, insertion, égalité des chances et dans la mesure où l'organisation de la journée demain le permet, en accord avec la commission des finances, nous pourrions porter exceptionnellement la durée maximale prévisionnelles sur cette mission de 2 heures 30 à 3 heures 30, y a-t-il des oppositions. Il y en a pas, il aurait ainsi décidé, je vais suspendre et la Suisse, la séance sera reprise à 14 heures 15 pour la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation, la séance est suspendue.